Dans quelles conditions la privatisation a-t-elle été réalisée ? Comment les tarifs sont-ils fixés ? Comment les nombreux avenants ont-ils été négociés ? Doit-on, en somme, mettre fin aux concessions ? C'est pour apporter un éclairage documenté et objectif sur ces questions récurrentes dans le débat public que la commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider a été créée sur l'initiative du groupe Union Centriste. Il s'agissait, d'une part, de faire la lumière sur l'idée selon laquelle l'État serait, en quelque sorte, floué par les concessions en cours au profit des groupes concessionnaires et, d'autre part, d'anticiper la fin des concessions, qui interviendra dans dix ans pour les premières, ainsi que de formuler des propositions cohérentes et équilibrées pour que la répartition des profits futurs soit juste pour l'État, les usagers et les exploitants. Tout au long de nos travaux, nous nous sommes donc attachés à analyser les relations entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes, et à retracer l'historique de la mise en place du réseau autoroutier. Nous avons, par ailleurs, cherché à évaluer de manière rigoureuse le niveau réel de rentabilité de l'exploitation des autoroutes. Enfin, nous nous sommes penchés sur l'effectivité des contrôles de l'État quant au respect des contrats en cours avec les concessionnaires. Les autoroutes sont un bien commun. Elles constituent des infrastructures de grande ampleur et un outil d'aménagement du territoire. Pour réaliser de longs trajets en voiture, nos concitoyens sont quasiment obligés de les parcourir. On peut donc considérer qu'il s'agit à la fois d'un service public et d'un monopole économique. Était-il dès lors souhaitable de la part de l'État de les privatiser ? Lorsque le Premier ministre Dominique de Villepin a décidé, en 2006, de privatiser les autoroutes, des ouvertures partielles du capital avaient déjà été réalisées depuis 2002. La situation budgétaire des SCA ne nécessitait pas d'intervenir en urgence et la majorité était d'ailleurs divisée sur le sujet- les auditions que nous avons menées nous l'ont confirmé. Le choix qui a été fait à l'époque a été de récupérer en une fois un montant élevé- 14,8 milliards d'euros - pour réduire la dette de l'État et financer de nouvelles infrastructures. Il s'agissait alors d'une décision politique. L'autre option était de continuer à percevoir, année après année, la rente que constitue l'exploitation des autoroutes, en assumant les aléas économiques : niveau du trafic, coût des travaux d'entretien Il n'est pas question ici de refaire l'histoire, mais d'envisager l'avenir. Notre commission d'enquête a estimé que les concessions en cours étaient trop longues d'environ dix ans au-delà de 2022, les dividendes versés devraient atteindre 40 milliards d'euros, à comparer avec les coûts d'acquisition des sociétés. Il apparaît donc impensable de prolonger les concessions en cours et si le choix est fait de les renouveler, lorsqu'elles arriveront à échéance, il faudra en réduire la durée. Je n'entrerai pas dans le détail de nos conclusions, car je vais laisser mon collègue rapporteur Vincent Delahaye s'en charger. Je souhaite simplement dire que le but du débat que nous avons aujourd'hui est de faire vivre le travail que nous avons mené. Nous ne voulons pas que notre rapport termine, comme bien d'autres avant lui, au fond d'un tiroir. Dès maintenant, nous devons préparer la fin des concessions et faire valoir notre rôle de parlementaires, qui consiste à peser dans la décision publique sur un sujet d'intérêt général. La parole est à M.

d'entretien et de maintenance. Il convient aussi de réfléchir à des clauses visant à un meilleur équilibre des contrats de concession- revoyure et partage des gains -et impliquer les usagers, à travers leurs associations, sans oublier le Parlement.

Mais tous les Français ont une expérience de l'autoroute. C'est parce qu'elles sont si ancrées dans leur vie, si indispensables à leurs déplacements, si structurantes pour nos territoires, qu'elles méritent toute notre attention. Elles méritent plus que des raccourcis et des débats simplistes. Il faut d'abord le rappeler, nos autoroutes sont un modèle de modernité, de confort et de sécurité. Oui, la France peut se targuer d'avoir l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur réseau autoroutier du monde.

depuis, le monde a changé et nos besoins aussi. Le paysage des acteurs autoroutiers, leur relation avec l'État et les contrats de concession sont bien différents de ceux qui prévalaient alors. Les contrats actuels, justement, doivent prendre fin de 2031 à 2036. C'est l'occasion de faire un bilan critique de notre modèle de financement et de gestion des infrastructures, sans complaisance ni démagogie. C'est l'occasion de le changer en mieux, de se demander quel est le modèle que nous voulons. Le Sénat s'est de nouveau saisi de cette question l'an passé en lançant une commission d'enquête sur les concessions autoroutières, dont M. Jeansannetas était président et M. Delahaye rapporteur. Je tiens à souligner la qualité de ses travaux et la pertinence d'une grande partie des analyses de son rapport. fournit des éléments d'éclairage précieux, tant sur les modalités d'amélioration des clauses contractuelles que sur les perspectives d'évolution du pilotage des contrats pour les années à venir. Nous avons examiné ses propositions avec attention et nous partageons un grand nombre de ses trente-huit recommandations. Pour preuve, près de 60 % d'entre elles sont déjà appliquées ou en cours de mise en oeuvre. car il y a un « mais » -nous avons un point de divergence, voire de désaccord, qui concerne vos estimations de rentabilité des concessions. Nous avons d'abord relevé des biais méthodologiques, puisque l'analyse s'écarte de la doctrine retenue par le régulateur, dont les équipes d'experts travaillent depuis six ans sur la question. Il y a aussi des écarts dans les projections. Certes, le sujet est complexe en cette période d'incertitudes liées à la crise sanitaire, mais entre la réalité des comptes des sociétés et les chiffres proposés par votre analyste, on passe du simple au double, voire du simple au triple Les résultats sont, là aussi, très éloignés de ceux du rapport quinquennal de l'Autorité de régulation des transports. Enfin, je regrette que le rapport installe une fausse polémique sur la question du plan de relance autoroutier entériné par le protocole de 2015, dont l'équilibre économique a pourtant été expressément validé par la Commission européenne, laquelle n'est pas spécialement laxiste sur ces sujets ! En d'autres termes, comme chaque fois qu'un rapport a été produit sur les concessions autoroutières, il n'existe aucun calcul ni aucune analyse qui prouverait de manière robuste une « sur-rentabilité » des sociétés concessionnaires. Plutôt que d'entrer dans cette polémique qui ne fait pas progresser le débat, il me paraît plus utile de concentrer l'action de l'État sur deux priorités : un meilleur encadrement des contrats et la projection de l'avenir du modèle des concessions.

Un dispositif limitant les éventualités de surprofits a été introduit dans les contrats historiques : en cas de surprofit, les tarifs de péages sont revus à la baisse ou la durée de la concession est réduite. L'État récupère toutes les économies faites par les SCA sur les investissements résultant des décalages de calendrier ou des abandons de projets. Le Parlement a également vu ses moyens de contrôle, d'évaluation et d'information considérablement renforcés. C'est ainsi au législateur qu'il revient d'autoriser l'allongement de la durée des contrats de concession. Les pénalités en cas de défaillance d'une société sur la sécurité, la performance ou l'état du réseau sont continûment renforcées. Enfin, la loi du 6 août 2015 a créé une autorité de régulation indépendante régulation des transports (ART), rend des avis publics sur les projets de nouveaux contrats de concession, mais aussi sur tous les projets d'avenants ayant une incidence sur les tarifs de péage. Elle produit annuellement une synthèse des comptes des sociétés concessionnaires et tous les cinq ans un rapport sur la rentabilité des contrats. Le premier rapport quinquennal de l'autorité a ainsi été publié à la fin de juillet 2020. Certes, les contrats historiques représentent la majorité du réseau, mais l'État a aussi passé de nouveaux contrats de concessions bien plus stricts. Tous ceux qui ont été passés depuis les années 2000 respectent globalement les recommandations de votre rapport. Notre deuxième priorité est de nous projeter, d'anticiper et de réfléchir à l'avenir des contrats de concessions. Je l'avais déjà rappelé en tant que député, je reste constant sur la question : l'enjeu principal est de penser à ce que nous en ferons demain de nos concessions.

Faut-il, à l'inverse, les prolonger ? Je sais que certains d'entre vous y sont favorables. Je sais qu'intégrer de nouveaux projets locaux par adossement pourrait être intéressant pour certains territoires, le cadre européen étant, là aussi, particulièrement strict. Mais je le disais, le monde a changé et nos besoins aussi. À trop vouloir prolonger les contrats du passé, nous risquerions d'accroître leur déconnexion avec les attentes des Français. Assurément, les contrats anciens doivent être modernisés.

Je n'ai pas de vision arrêtée ou dogmatique sur le sujet. Ma conviction est que nous ne devons pas brider nos réflexions : nous avons eu l'occasion au cours des débats en commission d'évoquer les concessions multimodales, les concessions régionalisées, les tarifs segmentés. Bref, un nouveau

En plus de cela, sur la même période, elles ont investi 20 milliards d'euros dans le patrimoine autoroutier. Sans le modèle concessif, des dizaines de projets d'infrastructures, au service des Français, n'auraient pu voir le jour. Pour aborder toutes ces questions et définir les aménagements à réaliser d'ici là, vous plaidez, monsieur le rapporteur, pour l'organisation d'un sommet des autoroutes. Sur le principe, j'y suis favorable. Il doit nous permettre de trouver comment gérer la « fin de vie » des contrats, sans les plonger dès maintenant dans un coma artificiel. Il me semblerait en effet insoutenable de ne procéder à aucun aménagement complémentaire dans les dix à quinze prochaines années. Nous avons déjà commencé à y travailler, en intégrant le déploiement de bornes électriques, les nouvelles mobilités ou l'expérimentation de péages en flux libre. Par ailleurs, nous avons besoin d'un cénacle où débattre des perspectives de gestion du réseau concédé. ces débats aujourd'hui et je m'engage à ce que nous puissions les poursuivre dans un horizon qui reste à définir. Le Parlement sera évidemment associé à ces réflexions. Mesdames, messieurs les sénateurs, cette question

Nos autoroutes doivent rester un atout pour la France, pour les Français, pour leurs déplacements. Elles doivent, mieux qu'avant, embrasser les enjeux écologiques et sociaux de notre temps. Nous allons maintenant Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires à condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

Christine Lavarde. Monsieur le ministre, les travaux de la commission d'enquête ont montré que la rentabilité pour les actionnaires serait atteinte autour de 2022. J'entends que vous contestez ces chiffres.

à rééquilibrer le partage de cette sur-rentabilité. Le Gouvernement va-t-il donner à l'ART les moyens de collecter auprès des sociétés d'autoroutes les informations nécessaires à l'analyse des variations de la rentabilité depuis 2002 ? Le Gouvernement va-t-il soutenir la proposition de loi déposée par le président du groupe Les Républicains,

des sociétés historiques, puisque c'est souvent à elles que l'on fait référence, sont estimées autour de 7,8 %, dans une fourchette oscillant entre 6,4 % et 9,2 %. Il est aussi indiqué que les taux de rentabilité interne ont enregistré une évolution favorable, mais modérée depuis 2007 le savez, le plan de relance autoroutier de 2015 n'a pas engendré de surcompensation. Les investissements prévus, à hauteur de 3,2 milliards d'euros, ont essentiellement porté sur des élargissements de sections et sur la construction ou la modification d'échangeurs. L'équilibre de la compensation dans le plan de relance autoroutier a été confirmé, je le soulignais dans mon propos liminaire, par la commission lors de sa décision du 24 octobre dernier. C'est la sous-estimation du taux de rentabilité

contrats historiques, en cas de surperformance économique sur la période d'allongement du contrat soit les tarifs de péage sont revus à la baisse, soit la durée de la concession est réduite. Par ailleurs, le gain financier issu de tout décalage dans l'exécution des investissements par ces sociétés est également et intégralement restitué au concédant.

En 2015, alors membre du groupe de travail sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes, j'ai refusé de signer les conclusions présentées par ce groupe pour une raison simple. Le calcul virtuel de la rentabilité à l'instant par l'Autorité de la concurrence omettait deux éléments essentiels

Comme toujours on se pose la question de la fin des concessions et du retour de l'État dans la gestion des autoroutes. Le rapport d'enquête est clair : le rachat des concessions, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, s'élèverait à environ 50 milliards d'euros Outre le fait que nous traversons une crise majeure, qui demande des moyens financiers importants, j'identifie deux problèmes supplémentaires : celui des recettes et celui du risque de non-affectation à l'entretien de notre réseau, qui est l'un des meilleurs d'Europe. Rappelons que l'État, avant la privatisation, percevait une manne très faible de la part des sociétés publiques qui exploitaient ce réseau. La réflexion autour de contrats plus équilibrés me paraît ainsi être la proposition la plus juste.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, le verdissement de nos autoroutes est une nécessité qui, loin d'être nouvelle, s'impose aujourd'hui fermement. Il est essentiel que les concessionnaires encouragent les mobilités à faible empreinte carbone, mais sans reproduire les erreurs passées. Le soutien à des mobilités écologiquement vertueuses doit se faire sans contreparties financières supplémentaires, car personne ne contestera la rentabilité économique des sociétés d'autoroutes. Ce n'est pas faire du concession démagogique

d'euros d'ici à 2036. Voilà l'argument que le concédant doit avancer au cours de la prochaine négociation pour « verdir » les tarifs et orienter les investissements vers la décarbonation sans compensation nouvelle. La prise en compte des enjeux environnementaux doit être une obligation contractuelle. C'est le principe même de l'écoconditionnalité. Pour préparer l'avenir, il faut rééquilibrer les contrats en faveur de l'intérêt public. Il s'agit de définir concrètement la responsabilité sociale et environnementale des concessionnaires. Dans le prolongement de la loi d'orientation des mobilités, le déploiement des bornes de recharge électrique doit passer à la vitesse supérieure. L'aménagement de voies réservées au covoiturage et aux transports collectifs doit nettement progresser, et des incitations tarifaires significatives être proposées aux véhicules les plus vertueux, en particulier pour les poids lourds. Sur les tronçons autoroutiers publics, une réduction tarifaire importante est d'ores et déjà proposée aux véhicules électriques. Ma question est donc la suivante : comment amener les concessionnaires à un cahier des charges ambitieux de décarbonation pour garantir que ces acteurs incontournables prennent réellement en compte l'objectif de l'accord de Paris ?

plans de relance de 2015 et l'avenant de 2018, plus de 400 millions d'euros cumulés ont été consacrés à ces investissements, qui étaient à l'époque historiques : ils ont permis de réaliser des ouvrages protégeant la biodiversité, d'améliorer l'assainissement ou encore de supprimer des points noirs du bruit. Pour autant, vous avez raison de le dire, il faut aller plus loin. Des expérimentations sont aujourd'hui pleinement satisfaisantes : je pense notamment à celles sur les flux libres. Nous avons lancé, en lien avec les concessionnaires, un grand plan de déploiement des bornes de recharge électrique.

équilibré entre l'État et les sociétés concessionnaires dans cette grande transformation écologique que nous accompagnons aujourd'hui. L'ensemble des propositions que nous avons reçues, tout comme les débats que nous avons pu avoir avec les élus, intègrent pleinement la dimension

en termes de longueur du réseau. Symbole du modernisme des Trente Glorieuses, ce réseau, concédé à 90 % à des sociétés à capitaux privés, a perdu de sa superbe. En effet, notre parc autoroutier, s'il est nécessaire et performant pour nos usagers, doit se réinventer, notamment pour se conformer aux nouvelles exigences environnementales. Pour autant, nous sommes défavorables à la renationalisation de nos autoroutes.

mobilités. Des investissements importants pourraient être mis en place en faveur du covoiturage, des parkings relais et des transports collectifs. Le projet de loi Climat et résilience, que nous examinerons prochainement, sera un véhicule pertinent pour proposer ces nouvelles alternatives durables. Monsieur le ministre, comment comptez-vous accompagner les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour qu'elles puissent se conformer à ces exigences ? La parole est à M. le ministre

Dagbert. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le rapport de la commission d'enquête indique que les dividendes versés aux actionnaires des concessions autoroutières devraient atteindre 40 milliards d'euros au-delà de 2022, chiffre que vous contestez. La privatisation de 2006 dont vous et nous héritons aujourd'hui s'est donc faite au détriment des contribuables, des usagers des autoroutes concédées, mais aussi des usagers des autres infrastructures de transport et du désenclavement des territoires. Cette manne aurait pu servir à financer une bonne partie du réseau routier national non concédé, à désengorger certains axes, à entretenir et développer nos infrastructures ferroviaires et à assumer des investissements qui nous ont fait tant défaut ces dernières années. Dans son référé en date du 23 janvier 2019, la Cour des comptes a affirmé que les divers plans de relance autoroutiers décidés en faveur du réseau concédé présentaient un risque de surinvestissement qui contrastait « avec le sous-investissement constaté sur le réseau non concédé Aussi, j'adhère totalement à l'axe 3 du rapport de la commission qui vise à négocier une amélioration du service rendu aux usagers. La réflexion porte sur le verdissement des tarifs des péages, les véhicules les plus propres, les bornes de recharge électrique, auxquels j'aimerais inclure les points de ravitaillement en hydrogène. En outre, il serait souhaitable que les sociétés concessionnaires d'autoroutes contribuent davantage au financement des autres infrastructures de transport, comme cela avait été décidé timidement en 2015 après l'abandon de l'écotaxe poids lourds, qui a engendré un manque à gagner de plus de 500 millions d'euros par an pour l'Agence de financement comment le Gouvernement entend-il optimiser l'allocation des investissements dans les infrastructures de transport, en les réorientant prioritairement vers celles qui sont structurantes pour l'aménagement du territoire et en encourageant la transition écologique dans le domaine des transports ? La parole est à M. le ministre délégué.

le deuxième sujet que vous avez, à raison, abordé est le sous-investissement chronique qu'ont subi les réseaux dits secondaires ou le réseau non concédé s'agissant de la route. Or, depuis 2017 et de façon constante, nous avons progressivement, tant sur les

Mieux qu'un rapport, ces travaux constituent un point d'appui utile et étayé pour mener le combat permettant le retour d'un État stratège en matière d'infrastructures d'intérêt national et d'aménagement du territoire. Depuis de trop nombreuses années, ce scandale perdure sans que rien s'oppose aux mastodontes privés. Les sociétés concessionnaires sont de véritables machines à cash puisque, même en temps de crise, même en 2020, les dividendes s'élèvent à 2 milliards d'euros. Entre 2006 et 2019, ce sont 24 milliards d'euros qui ont été distribués. Un « pognon de dingue » qui aurait été plus utile à la solidarité nationale ... Pourtant, les pouvoirs publics ne sont pas démunis. Je souhaiterais attirer votre attention, monsieur le ministre, et avoir votre avis sur un point précis. Il s'agit des obligations reposant normalement sur le concessionnaire au titre de l'article L. 3131-5 du code de la commande publique relatif notamment à l'inventaire du patrimoine. ce rapport n'a jamais été remis à l'autorité concédante, donc à l'État. Comment justifier cette opacité ? Comment, dans ce cadre, travailler à une reprise des concessions ? Comment comprendre que l'État, encore une fois, ne fasse pas respecter ses droits, au nom de l'intérêt public ? Monsieur le ministre,

d'un entretien soigné et régulier, ce patrimoine se détériore sous l'action du trafic et des agressions naturelles et nécessite alors des travaux de régénération considérables. La rénovation et le renouvellement de ce patrimoine se planifient et requièrent des travaux s'étalant sur plusieurs années dont les concessionnaires ont la responsabilité. En amont des fins de concession, l'action du concédant, c'est-à-dire l'État, en matière de contrôle du patrimoine et de politique d'entretien doit s'intensifier- c'est la fameuse clause des sept ans -afin d'éviter qu'un sous-investissement ne se traduise par une dégradation du patrimoine en fin de contrat. Depuis plusieurs années, l'État élabore une stratégie et un plan d'action pour structurer et renforcer l'efficacité de son intervention dans ce domaine. Trois chantiers ont ainsi été engagés avec les concessionnaires. Il s'agit d'abord de dresser un inventaire du patrimoine autoroutier concédé, ensuite de définir les outils et les méthodes permettant de mieux connaître, contrôler et suivre l'état fonctionnel du patrimoine, et enfin d'établir le bon état cible de ce patrimoine en vue de la préparation de la fin de contrat. Comme je l'évoquais précédemment, cet inventaire a été réalisé pour les ponts de Tancarville et de Normandie qui arriveront à échéance en 2027 et pour lesquels les échanges et les expertises techniques entre concédant et concessionnaire se sont déroulés sur près de deux ans entre la fin de 2018 et la mi-2020. La discussion n'a pas encore été engagée sur les contrats historiques puisque la clause des sept ans s'appliquera, par définition, sept ans avant les échéances de 2031 à 2036. Je souhaite que mon ministère, qui dispose de compétences et de moyens propres, continue d'assurer ces missions, en s'appuyant le cas échéant sur les équipes techniques du Centre d'études

tout dans ce dossier est ubuesque, de la conclusion des contrats aux sous-délégations qui favorisent les ententes en passant par la définition du niveau des péages. Dans une étude de 2020, deux universitaires français rappellent l'illégalité des surcompensations ainsi que celle du décret de 1995 indexant les péages sur l'inflation. Ces dispositifs pourraient être considérés soit comme des aides d'État au sens du droit européen, soit comme contraires aux règles définies par le code monétaire et financier,

Les conclusions de la commission d'enquête doivent permettre de préparer l'avenir, et c'est sur ce point que je souhaite vous interroger, monsieur le ministre. À l'heure de la transition écologique, on peut regretter que notre pays soit en retard sur le passage au péage sans barrière, qu'il est coutume d'appeler « flux libre En effet, l'intérêt d'un tel modèle est d'abord écologique : un poids lourd consomme deux litres de carburant supplémentaires en s'arrêtant et en redémarrant aux barrières de péage. Et ce sont de surcroît autant de surfaces imperméabilisées qui pourront être rendues à la nature. Monsieur le ministre, quels objectifs relatifs à ce modèle de péage du futur ont été fixés aux concessions autoroutières ? Dans un second temps, comme vous le savez, de nombreux poids lourds en transit évitent les autoroutes et empruntent des itinéraires parallèles les routes nationales ou départementales en raison de leur gratuité. Or la surfréquentation induite par une telle pratique pose des problèmes de sécurité parfois dramatiques, de dégradation évidente des infrastructures ou encore de nuisances sonores, sans parler d'une pollution de l'air accrue, quand les autoroutes sont mieux adaptées pour accueillir ces poids lourds. Alors qu'une mission d'information créée sur l'initiative de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable doit prochainement rendre ses conclusions sur le transport de marchandises face aux impératifs environnementaux, quelles sont vos propositions pour éviter ce report de trafic sur le réseau secondaire ? Pourquoi ne pas imaginer un dispositif sur le modèle des zones à faibles émissions pour les poids lourds ? Pensez-vous qu'il faille

C'est une demande des régions, notamment du Grand Est et de l'Île-de-France, à laquelle nous avons répondu. Les départements pourront également demander à l'appliquer sur certaines routes départementales pour éviter les reports de trafic. Les équipes de mon ministère travaillent actuellement à l'inventaire de ces routes au vu des demandes actuelles des élus.

J'ai deux questions sur ce sujet passionnant. Je salue la qualité des travaux de notre commission d'enquête, qui a bien mis en évidence un certain nombre de déséquilibres existant entre concédant et concessionnaires. Ma première question est courte le décret de 1995 relatif à la fixation annuelle du prix des péages est-il bien légal ? Dans l'hypothèse d'une abrogation, les conséquences seront importantes. Notre collègue députée Christine Pires Beaune attend toujours votre réponse à ses questions écrites : je ne doute pas que je vais l'obtenir. Ma deuxième question vient d'être posée par mon collègue Éric Bocquet. Elle est relative à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique doit publier chaque année un rapport contenant un inventaire précis et actualisé des biens concédés. Or cette obligation n'est pas respectée. Pis, monsieur le ministre, dans votre courrier du 5 avril adressé au rapporteur, vous écrivez que « l'enjeu pour le concédant n'est pas de disposer au cours de la concession d'un inventaire précis à un instant donné ». Cette phrase est totalement contraire à la doctrine législative et réglementaire. Vous n'avez pas répondu à mon collègue et ami Éric Bocquet, mais je ne doute pas que j'obtiendrai une réponse. Vous avez commencé votre propos introductif en déclarant que vous vouliez un meilleur encadrement des contrats. Pourtant, sur cette question qui n'est pas que technique, on donne les clés au concessionnaire et on ne le contrôle pas.

monsieur le sénateur, car je vous sais expert sur ces sujets. Sur l'abrogation du décret de 1995 d'abord, vous savez qu'il est prévu, par dérogation dispositions du droit commun, que les rémunérations des cocontractants de l'État au titre des contrats de concession puissent être indexées sur le niveau général des prix. Les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de ces dispositifs établissent clairement qu'il s'agissait surtout de conforter juridiquement la pratique contractuelle de l'État et des sociétés concessionnaires de recours à un indice d'évolution plutôt favorable soit à l'État, soit aux usagers. En outre, cette modification du code monétaire et financier avait le mérite de donner une accroche législative au décret de 1995 sur les péages autoroutiers. Cette dérogation ne nécessite pas forcément de décret d'application pour ces contrats administratifs. Il n'existe donc aujourd'hui plus de motif qui justifierait de remettre en cause le décret de 1995. Sur le sujet du bon état des infrastructures en fin de concession, j'ai répondu à M. Bocquet la stratégie de l'État en la matière était de structurer et de renforcer son intervention. Il s'agit de définir les bons outils et les bonnes méthodes qui permettent d'abord de connaître, puis de contrôler et de suivre, l'état fonctionnel du patrimoine afin d'établir le bon état cible

en écho à l'urgence dans laquelle nous nous trouvons actuellement et qui s'insère dans l'axe 3 développé dans le rapport de la commission d'enquête, à savoir négocier une amélioration du service rendu aux usagers compte tenu de la rentabilité indiquée dans le rapport. En 1970, la France était confrontée à un défi de développement économique des territoires : il s'agissait alors de « rattraper notre retard en matière de desserte des territoires par le réseau autoroutier », et le gouvernement d'alors avait fait appel au secteur privé. Dans la Sarthe, ce fut un succès, et nous l'avons constaté depuis les années 1970 avec l'A11 et depuis une vingtaine d'années avec l'A28. Cinq branches d'autoroute irriguent notre département et ont largement contribué à sa- modeste ! -prospérité économique. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'urgence climatique et à l'impérieuse nécessité de décarboner le secteur des transports, mais il faut rappeler que la route assure en France 87 % des déplacements de personnes et 86 % du transport de marchandises. Par conséquent, décarboner le secteur des transports signifie tout simplement qu'il faut décarboner la route : c'est urgent et nous ne pouvons pas attendre encore dix ans pour agir. Il me semble que nous sommes confrontés là aux exigences de nécessité et d'utilité prévues par l'article L. 122-4 du code de la voirie routière et la jurisprudence y afférente.

quelque peu différents. L'objectif, dans les années 1970, était de désenclaver les territoires avec des réseaux qui étaient peu construits et d'offrir des infrastructures adaptées pour un transport rapide et sûr. Je crois que, de ce point de vue, le bilan est objectivement bon cinquante ans plus tard.

Jocelyne Guidez. Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur la question des péages périurbains et de l'injustice que leur existence induit. Je pense en particulier à certains péages de la région Île-de-France, comme celui de Saint-Arnoult qui fut l'un des symboles de la crise des « gilets jaunes », ou encore celui de Dourdan que je connais bien. Notre réseau autoroutier a été construit à une époque où le développement périurbain n'avait pas encore atteint son niveau actuel, et où le recours à l'autoroute pour les trajets quotidiens entre le domicile et le travail était rare. Depuis, l'économie de services, c'est-à-dire des emplois urbains, s'est considérablement développée. Paris comme sa petite couronne ont attiré de plus en plus de travailleurs, de plus en plus éloignés, en raison notamment de l'explosion des prix de l'immobilier. Résultat, ce qui était hier l'exception est devenu la norme. Des dizaines de milliers de Franciliens prennent quotidiennement l'autoroute pour aller travailler. Un grand nombre d'entre eux sont contraints de payer les péages périurbains à chaque trajet. Cette obligation de payer pour aller travailler ne touche pas nécessairement les plus aisés. Devant la commission d'enquête, Jean-Claude Lagron, président de l'association « A10 gratuite » dont je salue l'engagement, indiquait qu'un travailleur régulier déboursait 1 300 euros par an. Lorsqu'ils ne veulent, ou ne peuvent, pas supporter ce coût, les travailleurs pendulaires se reportent sur le réseau routier secondaire, ce qui n'est pas sans conséquence en matière d'accidentalité d'accidentalité et de congestion. Votre prédécesseur, Mme Borne, avait certes obtenu un geste des sociétés d'autoroutes : une réduction de 30 % pour plus de dix allers-retours par mois sur le même tronçon. Si l'intention était bonne, l'opération a été un échec. Sur un million d'automobilistes prévus, à peine 100 000 ont finalement souscrit l'abonnement. Les concessionnaires ont peu communiqué sur cette offre et le geste n'était pas suffisant. Monsieur le ministre, la réponse doit être plus ambitieuse. La suppression de certains péages urbains, en particulier celui de Dourdan, serait une réponse appropriée. Comme le soulignait la commission d'enquête, cela n'aboutirait d'ailleurs pas à remettre en cause l'équilibre économique et financier de la concession Cofiroute. Négocier cette gratuité sans contrepartie tarifaire répondrait à une demande légitime d'équité. La le ministre délégué. Madame la sénatrice, vous évoquiez au fond le sujet bien connu des péages périurbains, fruit de la densification des aires urbaines et de leur impact sur le quotidien de leurs usagers.

les tarifs des usagers effectuant plus de dix allers-retours par mois. Ce dispositif a connu un début de succès : 130 000 abonnements ont été répertoriés, avec une hausse significative de 60 % entre septembre 2019 et septembre 2020.

Nous ne pouvons que nous féliciter de la production de ce rapport, qui a permis de mettre en évidence un assez grand nombre de points qui attestent des conditions, pénalisantes pour l'État, de la rédaction des conventions de concession. Le rapport met en effet en évidence bien des insuffisances, observables au moment de la cession des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Il semble notamment que celle-ci n'ait été précédée ni d'une révision des contrats dits « historiques » ni d'une définition de l'équilibre économique et financier des concessions.

Au-delà de la perte des recettes résultant, pour l'État, de la privatisation et du déséquilibre financier de la gestion de ces concessions autoroutières au profit des entreprises attributaires, le rapport souligne aussi la permanence des disparités dans les relations entre les sociétés concessionnaires du réseau autoroutier et la puissance publique, au détriment de cette dernière. Cela étant dit, ces concessions ont été validées ; dont acte. En outre, la réaction et les mesures qui en ont découlé attestent que, d'un point de vue juridique, il serait hasardeux d'y mettre un terme de façon anticipée. Pour

Si le rapport de la commission d'enquête rappelle que les clauses introduites en 2015 ont pu rééquilibrer les rapports entre l'État et les nouvelles SCA, il souligne néanmoins que ces clauses restent pour le moins inopérantes pour les SCA historiques. Cette situation de défiance menace directement les projets d'investissement de ces sociétés et les éventuels partenariats avec l'État ce sont nos territoires et les usagers qui pâtissent le plus de cette situation. Six ans après ces négociations, vu le contenu du rapport de la commission d'enquête, il devient urgent de réunir tous les acteurs et de négocier des clauses solides et durables, en toute transparence.

pour restaurer la confiance entre l'État et ses partenaires, mais aussi celle des usagers et de tous ceux qui sont intéressés par l'aménagement du territoire. Ces infrastructures sont essentielles pour l'ensemble du territoire national et il me paraît important que nous soyons associés de très près

si les recommandations de l'ART ont permis, au cours des dernières années, d'éclaircir quelque peu les conditions d'attribution des sous-concessions par les SCA, quelques zones d'ombre subsistent. Des progrès ont été réalisés pour renforcer l'effectivité de la modération tarifaire sur le prix des carburants, mais la commission d'enquête préconise un renfort des contrôles des sous-concessions. Deux mesures nous semblent souhaitables. La première serait de prévoir explicitement que l'ART puisse collecter directement auprès des sous-concessionnaires toute information utile pour contrôler le respect des engagements des titulaires concernant la fixation des prix ou la durée des sous-concessions.

Ma première question, monsieur le ministre, est donc simple : comptez-vous appliquer ces deux recommandations ? En second lieu, la crise sanitaire a mis en lumière le rôle des aires de services au sein du réseau autoroutier. Ce sont les sous-concessionnaires qui, par exemple, ont accueilli les routiers, les commerciaux et les autres usagers pour que ces derniers puissent se restaurer, se reposer et bénéficier de structures de confort, notamment en ce qui concerne l'hygiène. La crise a toutefois causé des pertes importantes pour les magasins, la distribution de boissons chaudes et la restauration.

Pourtant, ces derniers refusent de compenser le manque à gagner des sous-concessionnaires par des mesures économiques significatives. Voici donc ma seconde question : est-il envisageable d'instaurer un mécanisme de solidarité exceptionnel entre concessionnaires et sous-concessionnaires, dans le contexte de la crise sanitaire ?

à des pénuries de services essentiels- je pense notamment aux douches, aux toilettes, aux services de restauration -et, tous ensemble, nous nous sommes mobilisés pour les rouvrir le plus rapidement possible. Cela avait permis la réouverture, au cours des jours suivants,

dont Picoty Autoroutes est membre, et ces réunions ont permis de définir les demandes et les contraintes de chaque secteur. Elles doivent maintenant permettre de faciliter les négociations contractuelles entre concessionnaires et sous-concessionnaires. J'ai bon espoir que cette situation s'assainira dans les semaines ou mois qui viennent.

Ce mode de financement présente un triple avantage : il ne coûte rien à l'État, rien aux collectivités locales, qui n'auraient de toute façon pas les moyens de le financer, et rien à l'usager, puisque le tronçon sera gratuit. Dans ce dossier, mon interrogation est grande sur notre capacité et notre volonté à dépasser les polémiques infondées et les dogmatismes archaïques, afin de regarder la vérité en face et de prendre les bonnes décisions. L'importance économique de la mise en oeuvre de ce projet de plus de 300 millions d'euros me semble s'intégrer parfaitement dans le plan de relance et l'aménagement de notre territoire. Nous pourrions partager la conviction que, pour sortir de la crise actuelle, aux conséquences terrifiantes pour les finances publiques, notre pays aura besoin de recourir à l'investissement privé, afin de faire aboutir des projets d'infrastructures, en particulier routières.

acté son adossement à la concession d'ASF, seule et unique solution pour son financement et donc sa réalisation

Ce projet est connu ; il a fait l'objet de nombreux échanges depuis de nombreuses années, mais la métropole de Montpellier a décidé de se désengager de son financement, demandant un adossement total à la concession autoroutière existante. Par conséquent,

général. La parole est à M. Patrick Chaize. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les concessions autoroutières ont fait l'objet d'une contractualisation entre l'État et des sociétés privées, en prenant en compte des prévisions de dépenses et de recettes sur la durée du contrat c'est d'ailleurs la règle de base de tout contrat concessif. La règle est également de faire en sorte que le risque soit assumé par l'entreprise privée. Néanmoins, nous avons pu regretter la pratique de l'adossement, qui a consisté à ajouter des investissements non prévus initialement au contrat, en les compensant par un allongement de la durée de la concession initiale. Ce principe a pour inconvénient majeur de transformer le contrat, pourtant très précis, en un sentiment de concession perpétuelle, difficilement explicable à nos concitoyens et de moins en moins acceptable par eux. Si les Si les extensions de réseau peuvent être mieux maîtrisées et faire l'objet de procédures spécifiques, certains autres investissements nécessaires ne peuvent pas être dissociés du contrat. Je pense notamment à l'intégration des évolutions technologiques, telles que le développement des véhicules électriques et l'impérieuse nécessité de disposer, sur le réseau autoroutier, de bornes de recharge rapide. Plus encore, comment pourra-t-on intégrer les investissements nécessaires au déploiement des véhicules connectés ? Outre le besoin de choix technologiques partagés entre tous les acteurs, le montant des investissements nécessaires est loin d'être négligeable. L'urgence est pourtant là ; il serait irresponsable de repousser au terme des contrats les décisions d'investissement correspondantes.

Jusqu'à présent, 95 % des spécifications françaises sont reprises à l'échelon européen, ce qui est une satisfaction ; nous sommes face à une « terre d'opportunités ». Ces projets sont mis en place dans le cadre des concessions actuelles, sans prolongation.

je suis, comme ma collègue Jocelyne Guidez, qui s'est exprimée précédemment, et le rapporteur de notre commission d'enquête, Vincent Delahaye, sénateur du département de l'Essonne, et notre présence commune dans l'hémicycle ne doit certainement rien au hasard. En effet, depuis de nombreuses années, nous militons pour la gratuité des tronçons franciliens des autoroutes A10 et A11. Le périmètre de notre action est certes limité, mais parfaitement caractéristique et solidaire d'une problématique de dimension nationale. Depuis près de vingt ans, de multiples études ont dressé un constat, souvent accablant, des rapports entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Pourtant, rien n'a bougé, ou presque. Heureusement, le rapport de cette commission d'enquête sénatoriale confirme avec pertinence une situation de plus en plus inacceptable et esquisse de potentielles réponses, car ce débat doit déboucher enfin sur des mesures significatives ans, dans les territoires périphériques franciliens, l'étalement urbain a provoqué un triplement de la population. Durant la même période, les investissements en transports collectifs ont été quasi exclusivement concentrés dans le coeur de l'agglomération.

De ce fait, les autoroutes périurbaines ont dorénavant un rôle structurant pour les déplacements du quotidien, notamment les trajets domicile-travail. Pourquoi, alors, ne pas supprimer les péages sur les tronçons concédés des autoroutes périurbaines, à commencer par les plus iniques d'entre eux, sur l'A10 et l'A11, en Île-de-France ? pour financer cette disposition, monsieur le ministre : l'application de la clause de plafonnement de la rentabilité des concessions, issue du protocole de 2015, mais jamais mise en oeuvre, et l'instauration d'une taxe sur les copieux dividendes versés par les sociétés concessionnaires. Que pensez-vous de ces deux propositions ?

Des pistes d'amélioration sont évidemment à étudier ; je ne suis pas en mesure de répondre à votre question aujourd'hui, mais nous continuerons ces débats. Ainsi, des améliorations doivent être envisagées quant au trafic des poids lourds, qui pourrait se reporter sur la voirie locale. Je l'ai également évoqué, la contribution poids lourd régionale, que nous proposons dans le cadre de l'article 32 du projet de loi Climat et résilience, permettrait aux départements de se saisir de la possibilité d'étendre la contribution aux axes départementaux sujets au report de trafic. Je crois savoir que cette possibilité est étudiée en Île-de-France. Par ailleurs, des aménagements sur les voiries départementales sont aussi envisageables pour améliorer la sécurité et la fluidité des circulations qui traversent les zones habitées. Sur tous ces sujets, je reste évidemment à votre disposition, monsieur le sénateur, pour échanger et trouver les voies d'un avenir plus ensoleillé.

les dividendes versés à leurs actionnaires dépassent amplement leur résultat net. La crise sanitaire ne les affecte que marginalement, puisque, entre 2019 et 2020

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, pour autant qu'il m'en souvienne, lorsque j'étais au collège et que j'apprenais les différentes règles de l'orthographe de notre belle langue, je me demandais souvent : « Mais pourquoi ? » Alors, je prenais mon courage à deux mains et je demandais à mon professeur : « Pourquoi dit-on le soleil et la lune alors qu'en allemand le soleil est un terme féminin et la lune un mot masculin ? » Mieux encore, je lui demandais pourquoi les mots « orgue », « délice »

En effet, une langue est la résultante d'un travail lent et laborieux, de son usage par ceux-là mêmes qui la pratiquent, l'idéalisent et la malmènent. Elle n'est pas créée théoriquement ; elle est l'osmose plus ou moins parfaite des usages. Une langue n'est pas un bloc de marbre froid. Elle est un corps, une glaise qui se modèle, se sculpte, se transforme, se patine au gré du temps et de ses évolutions. Je ne suis ni linguiste ni philosophe. Je suis un humble sénateur inspiré par le bon sens. Vous l'aurez compris, je veux dire ici qu'une langue n'est pas le fruit de revendications identitaires et partisanes animées par une forme de militantisme bien désuet. Alors, quand j'ai découvert, indépendamment de toute idéologie, le sujet de l'écriture inclusive, j'ai cru à une fantaisie, une sorte de caprice de l'esprit. Je vous le confie, tout cela me semblerait dérisoire s'il ne révélait pas l'expression d'une fracture de la société, raison pour laquelle notre groupe vous invite aujourd'hui à réfléchir sur l'écriture inclusive. Avant tout, revenons aux réponses, loin d'être satisfaisantes, de mon professeur. Nombre d'entre vous ont dû entendre les mêmes de la bouche de leurs enseignants. Pourtant, cela ne vous a pas empêchés d'acquérir les rudiments de l'orthographe française. Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux face à la langue. Je ne pense pas me tromper en observant une lente et pernicieuse dégradation de l'apprentissage de notre langue parmi les jeunes générations. Avant de s'intéresser à l'écriture inclusive, comme notre groupe vous y invite, commençons par apprendre la langue française à nos enfants ! Interrogez nos universitaires et nos enseignants : ils sont désespérés. Je veux vous lire le témoignage que j'ai recueilli auprès d'une professeure de faculté : « Mes étudiants comprennent un raisonnement, une démonstration, mais ils sont, pour la plupart, dans l'incapacité de retranscrire ce raisonnement, faute de savoir construire une phrase simple, avec un sujet, un verbe et un complément, voire, parfois, ne disposant que d'un vocabulaire d'une pauvreté abyssale. » Le linguiste Alain Bentolila corrobore ces propos avec un chiffre effrayant : « 20 % des jeunes possèdent moins de 500 mots pour dire le monde. Je crains que nous ne puissions parler de générations sacrifiées. Je présume que les nouvelles technologies, avec les « réseaux antisociaux », pour citer le président de notre groupe, Claude Malhuret, ne vont pas contribuer à améliorer les choses Même si notre ministre a décidé de réformer la pédagogie, il faudra des décennies pour rattraper le temps perdu et les dégâts occasionnés. Si les tentatives de pratique de l'écriture inclusive prêtent à sourire, cette vérité n'a rien d'amusant. Revenons à nos moutons et tentons de comprendre l'origine du phénomène de l'écriture inclusive. Le mouvement est d'origine anglo-saxonne et serait l'initiative d'associations féministes dénonçant une masculinisation à marche forcée de la langue française que l'invisibilité de l'appartenance sexuelle et, bien entendu, celle du sexe féminin. Le coeur de cette graphie se résume dans la mise en cause de la règle, datant du XVII siècle, selon laquelle « le masculin l'emporte sur le féminin ». Le grammairien et académicien Nicolas Beauzée précisait : « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin, à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » Bah voyons ! C'était en 1767 Vous le savez aussi bien que moi, mes chers collègues, l'écriture de l'histoire ne se regarde pas avec les yeux d'aujourd'hui, mais nous pouvons comprendre la colère que de tels jugements peuvent entraîner et tenter, à la demande de certains mouvements féministes, de corriger ce prétendu déséquilibre. Il n'est pas question d'interdire d'interroger l'orthographe. Toutefois, l'écriture inclusive ne s'arrête pas là. Si j'ai bien compris, elle consiste à insérer des points médians à la fin des noms pour féminiser l'écriture. Cette pratique, loin d'être intuitive, peine à s'imposer. En mars 2017, un premier ouvrage destiné à des élèves de CE2 en écriture inclusive a été publié. Certaines écoles ou universités et même des collectivités territoriales auraient également lancé des initiatives destinées à encourager cette écriture.

identificateurs de sexe : pour certains, la langue française a trouvé et trouve commode de détourner l'usage arbitraire des marques de genre pour obtenir une distinction entre les femmes et les hommes. On peut discuter des règles, tenter de les comprendre. Mais, je le répète, seuls l'usage et le temps font finalement évoluer notre langue. Cela me conduit à une réflexion

Quand je parle de cette graphie, on me regarde avec des yeux ronds, avant de balayer le sujet de la conversation pour se concentrer sur ce qui est important. Ce débat semble s'autoalimenter dans des sphères dites « bien-pensantes », politiquement correctes, aussi appelées, à l'américaine, « éveillées ». Cette graphie, plus qu'une réelle revendication, serait devenue une sorte de marqueur idéologique, un signe extérieur de richesse culturelle, la Rolex de la bien-pensance.

font preuve d'une remarquable homogénéité de pensée, de genre ou de pigmentation de la peau. Contrairement à ces derniers, je me refuse à parler de race ou même à réduire mes compatriotes à leur couleur de peau, leur genre ou leurs origines. Quand Jacques Derrida disait « je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne », il mettait en avant un caractère essentiel de la langue : le fait qu'elle n'appartient à personne, qu'elle n'est donc pas un outil idéologique La question de l'égalité entre les femmes et les hommes est, bien entendu, première. Dès lors, pourquoi ne pas poser cette question directement ? Reléguer la gent féminine à un « e » final séparé par un point ne serait-il pas aussi une manière de mettre un point, final cette fois, à la discussion ? J'y lis, entre les points, un violent renoncement à l'égalité. Je ne sais pas si je dois m'en offusquer ou m'en attrister. Il est dit que l'écriture inclusive consiste à inclure toutes les personnes pouvant ne pas se sentir représentées, sur le plan du genre, de l'ethnicité ou de la religion. la demande de certains groupes féministes, nous aurons à modifier notre langue sous la pression d'autres groupes de revendication ? Mes chers collègues, voulons-nous nourrir cette archipélisation de la société française qu'a si bien décrite Jérôme Fourquet et qui amène Jacques Julliard à observer « le passage de la République des citoyens à la société des individus », inspirée par certains courants outre-Atlantique, que certains exportent ici Nous ne pouvons pas admettre cette volonté d'asservir les droits de l'Homme au profit d'une dictature de minorités défendant des intérêts particuliers. Je n'ai pas oublié, pour ma part, que les valeurs qui nous animent sont les principes de République, de liberté, de 'égalité et de fraternité, quatre termes dont je ne revendique pas la masculinisation ! Ces valeurs sont trop précieuses, lumineuses et universelles.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'écriture inclusive alimente régulièrement les polémiques en se faisant l'écho d'un sujet sociétal majeur : l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour autant, l'écriture inclusive caricature ce combat et, à mon sens, porte plusieurs dérives, que je veux rappeler La première est issue d'un présupposé : la pratique de la langue doit être une déclinaison des politiques sociales inclusives, donc inclure toutes les personnes qui peuvent se sentir non représentées. La langue refléterait ainsi fidèlement l'ordre du monde, la façon de penser d'une société., une langue qui invisibilise le féminin au profit du masculin serait celle d'un monde où les femmes sont cachées. Aujourd'hui, l'écriture inclusive servirait donc les luttes féministes. Qu'en sera-t-il demain lorsque la langue devra servir une autre cause ? Faudra-t-il changer de langue au gré des combats sociétaux ? Erik Orsenna, dans, nous alerte sur les dangers de la confusion entre ordre linguistique et ordre social. Dans ce conte, il narre les aventures d'un dictateur qui, voulant lutter contre les bavardages pour hisser son pays au rang de puissance mondiale, bannit les mots inutiles. « Évidemment, c'était plus facile de déclarer la guerre aux mots que d'affronter le chômage ! », déclare son héroïne deuxième dérive de l'écriture inclusive est sa vision de la masculinité dans le langage. Comme nombre d'entre vous, j'ai appris, dans les leçons de grammaire, que « le masculin l'emporte sur le féminin ». Cette règle concentre les attaques des partisans de l'écriture inclusive. Toutefois, les linguistes déconstruisent la thèse selon laquelle elle aurait été instaurée afin de soumettre les femmes. Depuis la première moitié du XVII siècle,

En fait, le masculin fonctionne en français comme le genre de base, portant la généralité. C'est au masculin qu'est formé le participe dans « j'ai écrit »,

multiplication des lettres muettes, la révision de la ponctuation, la complexité des règles d'accord, la fin de la linéarité de la chaîne écrite autant de difficultés nouvelles qui entraînent une perte de compréhension. Quel en sera le coût social ? Quels en seront les bénéfices ? Surtout, quels en seront les bénéficiaires ? lorsque l'on nous dit que l'écriture inclusive n'a pas vocation à être imposée aux écoliers, en particulier à ceux qui éprouvent des difficultés à entrer dans l'écrit, n'est-on pas à même de s'interroger sur la prétendue inclusivité de l'écriture inclusive ? Pour ma part, je crois profondément que l'écriture inclusive ne répondra pas aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes. Au contraire, elle créera un fossé entre ceux qui la maîtrisent et ceux qui n'auront pas accès à cette complexité coupée du monde réel. La langue est un vecteur de partage et de rassemblement. J'en veux pour preuve le rôle joué par notre école depuis près de cent cinquante ans, qui a permis à des enfants non francophones arrivés en France de parler français et, ainsi, de s'intégrer dans notre société et de faire Nation. La langue est bien l'un des facteurs premiers d'intégration. En août 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, en rendant obligatoire l'usage du français dans les actes publics de justice et d'administration du royaume, précisait que les arrêts devaient être clairs et compréhensibles, afin qu'il n'y ait pas de raison de douter sur leur sens. Dans une langue, les objectifs de clarté et de compréhension sont des défis perpétuels. Ils le sont particulièrement aujourd'hui. Il me paraît dangereux de sacrifier l'apprentissage de l'écriture et de la lecture sur l'autel de l'instrumentalisation de notre langue à des fins idéologiques. Sans fondement historique, sans pertinence linguistique, loin d'être inclusive, cette écriture est, au contraire, facteur d'exclusion entre ceux qui maîtrisent et ceux qui subissent. Ni notre langue ni notre société n'en ont besoin.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, chers collègues, l'idée selon laquelle le pouvoir des hommes et, en l'occurrence, le pouvoir des femmes se refléteraient dans le choix des mots n'est pas nouvelle. La volonté de réformer une langue pour marquer un changement sociétal ne l'est pas non plus. Jamais la langue française n'aura connu autant de changements que sous la Révolution française. Le français a été érigé comme langue nationale, arme défensive pour prémunir la République de tout morcellement. Trait d'union entre tous les citoyens, elle a contribué à cimenter l'identité républicaine, en offrant à chacun un égal accès aux lois, au droit, à l'instruction. Dans le même temps, le français s'est considérablement enrichi et n'a jamais cessé de le faire, en intégrant des mots en patois, des mots étrangers, des innovations lexicales. La langue française est avant tout une langue vivante, à la fois chargée d'histoire et évolutive. L'écriture inclusive a déjà imprimé son empreinte à travers la féminisation des métiers et des fonctions, la suppression du « mademoiselle » dans les documents administratifs ou encore le choix spontané de certains mots neutres pour inclure l'ensemble des interlocuteurs, comme je l'ai d'ailleurs fait au début de mon discours en préférant le mot « collègues » à « sénateurs » ou « sénatrices et sénateurs En la matière, le mieux est l'ennemi du bien, et il ne faudrait pas confondre les évolutions naturelles de la langue, partagées par la majorité des Français, et sa confiscation par une petite minorité porteuse de revendications égalitaristes. Cette offensive lexicale se cristallise dans l'usage du point médian, qu'une poignée de militants tentent d'imposer dans les universités, certaines mairies ou dans les écoles. Cette écriture prétendument inclusive se révèle en pratique inaccessible pour un grand nombre de nos concitoyens,

Les témoignages que nous avons recueillis soulignent que, en modifiant la graphie des phrases, l'écriture inclusive rend les textes absolument incompréhensibles pour toute personne qui utilise la lecture d'écran par synthèse vocale. En cherchant à dégenrer la langue, nous fabriquons une langue d'exclusion, une langue discriminante. Nous devons faire usage de bon sens et veiller par-dessus tout à l'accessibilité de la langue pour tous, avant de chercher à la rendre conforme à nos revendications idéologiques, justifiées ou non. À l'heure où nous débattons de la symbolique des mots, des millions de femmes dans le monde sont prisonnières de sociétés profondément machistes, sexistes et violentes à leur égard. Alors que certains se hérissent au nom de la théorie du genre, des femmes sont lapidées, brûlées à l'acide au nom de la tradition ou pour avoir refusé une demande en mariage. Il faut choisir ses combats, ceux qui en valent la peine. La journaliste d'origine turque, Claire Koç, a choisi la France précisément pour les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité que notre pays incarne et défend. Je dis bien « fraternité », mot féminin qui désigne le lien existant entre les membres de la famille humaine, que les mêmes défenseurs du point médian voudraient doubler du mot « sororité », quitte à modifier la devise républicaine au nom d'un faux féminisme revanchard. La différence, c'est que la sororité n'inclut pas les hommes, alors que la fraternité inclut les femmes et les hommes. La galanterie est-elle toujours permise ou allons-nous bientôt chercher à en faire une marque de sexisme insupportable ? L'historienne Mona Ozouf plaide pour l'apprentissage de la nuance et défend l'idée qu'il existe un féminisme à la française, où la galanterie reste l'expression d'une élégance. Vous l'aurez compris, chers collègues, je suis pour une société inclusive et une langue française universelle, qui facilite qui facilite la lecture et la compréhension. C'est la raison pour laquelle je suis contre cette écriture d'exclusion que représente l'usage du point médian. La

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens à remercier le groupe Les Indépendants - République et Territoires de nous avoir proposé ce débat, d'une importance capitale pour traiter d'un péril civilisationnel aussi majeur que l'écriture inclusive, ou, plus exactement, le terrifiant point médian. Malgré la pandémie, l'explosion des inégalités, la crise sociale, malgré l'effondrement de la biodiversité et la catastrophe climatique qui s'annoncent, vous avez su garder la tête froide et remettre au coeur de la Haute Assemblée les vrais débats qui comptent. Cela doit être salué. Puisque nous devons débattre, faisons-le sérieusement. La langue est une construction culturelle et sociale. et sociale. Elle reflète notamment les évolutions et les rapports de force dans la société. À son tour, elle forge les esprits : elle détermine en partie la manière dont nous pensons et envisageons le réel. Le langage porte en lui des questions politiques. Il est forcément l'objet d'évolutions et de tensions. L'écriture inclusive, ou plutôt le souci d'une communication inclusive, est une forme de travail sur ce langage. C'est un processus de réappropriation de la langue, pour plus d'égalité. En France, ce débat s'est focalisé sur le point médian, comme nous le voyons aujourd'hui. Pourtant, celui-ci n'est pas l'alpha et l'oméga d'une communication inclusive. Bravo ! Mais le niveau de débat actuel, qui ne permet aucune nuance ou réflexion, passe désormais par un processus bien rodé : des personnes, des chercheuses ou des militantes, réfléchissent sur un sujet, font une proposition, qui rompt parfois avec une forme d'ordre établi ; puis, les réactionnaires ou les conservateurs, paniqués par toute forme de progrès, montent le sujet en épingle pour nier l'exigence d'égalité. Les polémiques se cristallisent sur de faux problèmes et l'on finit par disserter ici sur de la typographie. Oui, nous pouvons questionner notre communication, y compris dans nos administrations, quand elle invisibilise parfois 50 % de la population ! Non, le point médian, celui qui coupe les mots pour leur ajouter un suffixe, n'est pas le seul outil d'écriture inclusive ! Non, ce n'est ni un « péril mortel » ni un « risque civilisationnel lire ! Comment diminuer les inégalités qui se trouvent au coeur même de notre manière de nous exprimer, donc de rendre compte du réel ? La langue française est une langue vivante. Elle évolue avec les femmes et les hommes qui la parlent. Il en a toujours été ainsi. Il serait illusoire de vouloir inscrire dans le marbre des règles immuables et de fixer définitivement les usages. Les seules langues ainsi figées sont les langues mortes, comme le grec ou le latin. J'espère que personne ici n'a cette ambition pour notre langue nationale. Parmi les arguments souvent cités à l'encontre du point médian, nous venons de l'entendre, un argument revient sans cesse, qui s'avère tout à fait exact : son usage rend la lecture difficile pour les personnes souffrant d'un handicap de lecture. C'est même en raison de cette difficulté que Jean-Michel Blanquer souhaite interdire son usage à l'école. C'est le bal des tartuffes ! Cette soudaine passion pour les enfants en situation de handicap disparaît soudainement quand il s'agit de revaloriser le salaire des accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH, qui sont mobilisés depuis des mois pour la reconnaissance de leurs missions. Au-delà du point médian, le fond du problème est la prédominance du masculin dans notre langue. Cela s'explique par l'histoire, par une évolution lente, depuis un latin qui reconnaissait trois genres- féminin, masculin et neutre -jusqu'à la progressive disparition du genre neutre au profit d'un masculin qui devint générique.

Même lors de la fondation de l'Académie française par Richelieu et alors que les règles que nous connaissons aujourd'hui se sont stratifiées peu à peu, la règle de prédominance du masculin n'a jamais été aussi fortement affirmée qu'elle ne l'est aujourd'hui. On préférait ainsi, par exemple, l'accord de proximité, qui consiste à accorder le genre de l'adjectif avec le nom le plus proche qu'il qualifie. Mes chers collègues, sachez ainsi que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, je le rappelle, a valeur constitutionnelle, mentionne : « Tous les Citoyens [ ...] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics.

côté, aux prétendus délires séparatistes d'une partie de la population. Il s'agit d'un processus d'évolution de la langue, nourri par un questionnement. Ce processus interroge et nous élève. Oui, il est possible de communiquer en incluant toute la diversité de notre société ! Non, vous n'êtes pas et vous ne serez jamais obligés d'utiliser le point médian ! Notre langue est riche quand elle se réinvente. Soyez donc inventives et inventifs ! Pour conclure, je tiens à faire remarquer à cette assemblée que le discours que je viens de prononcer, comme tous ceux que prononcent les sénatrices et sénateurs de mon groupe, a été réalisé en suivant dans la mesure du possible les règles de cette langue épicène que vous fustigez tant. Chacun sera libre de constater si celui-ci a mis en danger la langue française ! La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, inscrit à l'article 1 de notre Constitution, est une juste cause. Il mérite une action résolue, ambitieuse et ininterrompue. En parallèle, l'article 2 de notre Constitution dispose que « la langue de la République est le français ». Il s'agit d'un facteur d'intégration, d'appartenance et de rayonnement de la culture française. Notre langue nationale constitue le socle fondamental de notre fraternité républicaine. Le débat sur l'écriture épicène, dite « inclusive », met en jeu ces deux exigences constitutionnelles. Au-delà, elle interroge notre façon de « faire société » à travers le langage. L'écriture inclusive repose sur deux grands principes. D'une part, il s'agit d'accorder les grades, fonctions, métiers et titres en fonction du genre- on écrira ainsi « une autrice », « une pompière une sénatrice ». Ce principe ne rencontre pas d'opposition, et l'Académie française en a d'ailleurs fait la promotion. Il s'agit de lutter contre l'invisibilisation des femmes. D'autre part, il s'agit d'inclure les deux sexes grâce à l'utilisation du point médian pour éviter que le masculin « ne l'emporte » sur le féminin- on écrira ainsi « les électeur.rice.s » ou « les citoyen.ne.s C'est ce principe qui attise aujourd'hui les passions. Albert Camus disait : « J'ai une patrie : la langue française. » Or non seulement l'écriture inclusive conduit à une dénaturation de la langue française, mais le désir d'égalité n'excuse pas le façonnage des consciences. Cette écriture s'accompagne en effet d'une politisation du langage de la part d'une minorité loin d'être consensuelle. Elle n'est utilisée que dans des cercles militants très restreints, et sa généralisation semble au moins prématurée, au pire peu souhaitable. Comme notre collègue Bargeton, Roland Barthes : « Dès qu'elle est proférée, fût-ce dans l'intimité la plus profonde du sujet, la langue entre au service d'un pouvoir. » Oui, la langue entre au service d'un pouvoir, celui de la culture et de l'histoire dont nous sommes héritiers Le français est riche d'un passé glorieux. Nos écrivains, nos diplomates, nos figures illustres ont pensé dans cette langue prestigieuse dont l'influence est forte dans les pays de la francophonie. Mais la langue française ne doit pas être instrumentalisée au service d'une repentance anachronique. L'écriture inclusive relève d'une idéologie militante dont ne doivent pas souffrir les élèves. Alors que ces derniers ont de plus en plus de mal à savoir lire et écrire, comme nous le démontrent les classements PISA, nous ne pouvons nous permettre d'alourdir et de complexifier l'apprentissage de la langue française. L'Académie française a déjà alerté sur le risque d'aboutir à une langue désunie, disparate dans son expression et créant une confusion qui confine à l'illisibilité. Très bien ! L'écriture inclusive consacre une rupture sans précédent entre la langue parlée et la langue écrite. Si chacun est libre d'utiliser divers moyens de communication dans son espace privé, les services publics, ainsi que leurs agents, ne doivent pas communiquer par écrit dans une langue aussi incomprise que discriminante. À cet égard, je ne peux que soutenir la décision du ministre de l'éducation nationale de rejeter l'usage de l'écriture inclusive dans les manuels scolaires. Il s'agit d'un barrage à la transmission de notre langue pour tous, raison pour laquelle je m'inscris en opposition, ainsi que l'ensemble de mon groupe, avec cette écriture compliquée. Loin de tout discours réactionnaire, je ne peux me résoudre à lire un « roman épicène »- de grâce, épargnez-moi l'allongement des fameuses phrases de Proust !

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mesdames les sénatrices, mesdames les sénateurs, messieurs les sénateurs, chères collègues,

Vous avez reconnu, chers collègues, l'une des prescriptions de l'ordonnance sur le fait de la justice, prise en 1539, à Villers-Cotterêts, par François I en un château où il reçut François Rabelais et Clément Marot. Quatre siècles plus tard, l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 déclare toujours que « la langue de la République est le français », mais, pas plus que l'ordonnance de 1539, la Constitution ne précise de quel français il s'agit. Toutefois, dans sa sagesse, le procureur général du roi avait précisé, en 1539, qu'il s'agissait du français comme langue maternelle, c'est-à-dire de la langue telle qu'elle est parlée dans la diversité de ses pratiques, de ses emprunts et de ses assimilations. Cette langue a beaucoup évolué depuis le XVI siècle, et ses transformations successives ont accompagné celles de nos sociétés pour qu'elle demeure, en ce début du XXI siècle, « ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre Dans le monde, le français est aujourd'hui la langue de près de 300 millions de personnes, qui l'utilisent, la font évoluer et l'adaptent à des réalités sociales en perpétuelles mutations. Ces locuteurs, peut-être parce qu'ils ont une relation avec la langue française moins sacramentelle que la nôtre, lui apportent beaucoup pour qu'elle demeure vivante. Ainsi, le 28 juillet 1979, la publiait une publiait une instruction de l'Office de la langue française qui recommandait l'utilisation des formes féminines dans tous les cas possibles, soit à l'aide du féminin usité- une infirmière -, soit à l'aide du seul déterminant- la ministre -, soit par un néologisme- une chirurgienne -, soit par l'adjonction du mot femme : une femme-ingénieur. On sait qu'une circulaire gouvernementale du même esprit, proposée par Mme la ministre Yvette Roudy en 1986, suscita une vive réaction des geôliers de la langue, qui lui reprochèrent de vouloir « enjuponner le vocabulaire ». Pourtant, l'usage a tranché, et je note que notre assemblée compte quatre-vingt-dix femmes qui ont souhaité se faire appeler « sénatrices », alors que vingt-huit autres demandent qu'on leur donne du « sénateur ». En revanche, je n'ai pas trouvé d'homme revendiquant le titre de « sénatrice Cette liberté donnée à la pratique de la langue doit être préservée, car elle fait toute sa richesse. Je note, avec malice, que la direction de la séance de notre assemblée n'applique pas à la lettre les rectifications orthographiques du français recommandées par l'Académie française en 1990. Ainsi, dans nos comptes rendus, le mot « événement » garde fièrement ses deux accents aigus, alors que l'Académie préconise de changer le second par un accent grave.

S'agissant de l'utilisation typographique du point médian, il nous faut écouter un autre Conseil de la langue française, celui de la communauté francophone de Belgique, qui recommande un « emploi parcimonieux de ces formules » afin de ne pas trop entraver la lecture et l'écriture. Sans dénier tout intérêt à ce débat, nous eussions préféré qu'il portât plus largement sur le recul de l'emploi du français dans de nombreux domaines de nos activités. Je pense notamment à celui de la recherche, pour lequel les organismes nationaux obligent autoritairement leurs agents à publier dans un volapük vaguement dérivé de l'anglais. Pour la défense et illustration du français, il serait nécessaire, madame secrétaire d'État, que votre gouvernement appliquât la loi dite Toubon du 4 août 1994. C'est protéger et promouvoir avec intelligence le français impose de ne point figer son usage par des règles désuètes qui en réserveraient la pratique à une petite caste de scribes. Sur ce point, je conclus par cette citation d'Ernest Renan dont l'intelligence des relations d'une langue avec la Nation demeure d'une grande actualité : Les langues sont des formations historiques, qui indiquent peu de choses sur le sang de ceux qui les parlent. » Il ajoute qu'une considération exagérée donnée à la langue a ses dangers On se renferme dans une culture déterminée, tenue pour nationale ; on se limite, on se claquemure. On quitte le grand air qu'on respire dans le vaste champ de l'humanité pour s'enfermer dans des conventicules de compatriotes. »

sans que l'appellation correspondant à leur activité et à leur rôle réponde pleinement à cette situation nouvelle. L'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la reconnaissance du rôle de ces dernières dans la société est un combat juste, qui me tient particulièrement à coeur en tant que présidente de la délégation aux aux droits des femmes. L'écriture inclusive, dont nous débattons aujourd'hui, se présente comme un des outils permettant d'offrir une meilleure visibilité aux femmes. Par l'écriture inclusive, on entend un ensemble de pratiques et d'annotations qui vise à donner une représentation égale des femmes et des hommes dans la langue écrite. Mais devons-nous penser qu'une modification des règles grammaticales de la langue française écrite sera un moyen de parvenir à une égalité entre les femmes et les hommes ? Je ne le crois pas. Au-delà de l'objectif qu'elle poursuit, l'écriture inclusive pose plusieurs problèmes. Le premier est une réelle difficulté d'apprentissage : l'écriture inclusive rompt avec les règles de prononciation et de ponctuation, ainsi qu'avec les règles morphologiques que les jeunes élèves sont en train d'acquérir. De nombreuses associations de parents d'élèves ainsi qu'une large partie du corps enseignant se sont montrées hostiles à son application dans l'enseignement. Le ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, s'est d'ailleurs prononcé contre cette pratique dans l'éducation nationale en octobre 2017. Simultanément, l'Académie française alertait sur le risque d'aboutir à « une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l'illisibilité L'écriture inclusive pose ensuite un problème majeur pour les personnes souffrant de handicap, comme cela a déjà été souligné. Je pense, par exemple, aux personnes malvoyantes et aux élèves dyslexiques ou dyspraxiques. Pour les personnes malvoyantes, le problème est insoluble : tous les systèmes d'écriture connus ont vocation à être oralisés. Or il est impossible de lire l'écriture inclusive : « cher.e.s » ne se prononce pas. Le décalage graphie-phonie ne repose plus sur des conventions d'écriture, mais sur des règles morales que les programmes de synthèse vocale ne peuvent traiter et qui rendent les textes inaccessibles aux malvoyants. L'écriture inclusive devient donc, de fait, excluante pour une partie de la population. Elle se transforme en pratique complexe et élitiste. Offrir une meilleure visibilité aux femmes dans nos sociétés est un but à poursuivre avec force et détermination, il ne me semble pas que l'écriture inclusive soit le meilleur moyen d'y parvenir. Je ne crois pas qu'une mutation d'ordre syntaxique puisse permettre d'accélérer une mutation sociale. C'est le sort fait aux femmes et l'usage de la langue qui doivent évoluer et non la langue elle-même. Puisqu'il est question d'égalité au travers de ce débat, permettez-moi un hors sujet ayons une pensée pour Chahinez Boutaa et les trente-huit victimes de féminicides depuis le début de l'année. Ces crimes inqualifiables démontrent notre incapacité à protéger ces femmes. C'est le triste constat d'une société inégalitaire au sein de laquelle, en termes de violences subies, le féminin l'emporte sur le masculin. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, « ce qui n'est pas nommé n'existe pas », écrivait le poète turc Ilhan Berk. C'est incontestable : la langue que nous écrivons, que nous parlons, joue un rôle essentiel dans notre représentation du monde. Au cours des derniers siècles, elle a éludé, invisibilisé les femmes. Leur redonner leur juste place et ainsi ouvrir le champ des possibles, c'est tout le projet de l'écriture inclusive, que je préfère pour ma part qualifier d'écriture « égalitaire », et qui englobe en réalité un éventail de techniques. Je nous invite, pour avoir un débat constructif, à la regarder telle qu'elle est, loin de toute caricature : accord de proximité, féminisation des noms de métiers, titres et fonctions, dits « épicènes », formes féminines et masculines pour parler d'un public mixte- abrégées ou non par le recours au point médian ... Autant d'outils dont peuvent se saisir celles et ceux qui souhaitent encourager dans la langue une égalité de représentation entre les femmes et les hommes. Parmi ces techniques, c'est le point médian, dernier symbole d'une logique typographique visant à faire ressortir les formes féminines, qui polarise le plus les critiques. Ce point médian suscite des troubles, des inquiétudes, quant à son maniement et à sa lisibilité, y compris au sein de mon groupe. Ces doutes, je les entends d'autant plus qu'ils peuvent être alimentés par de mauvais usages. lorsqu'on pratique bien l'écriture inclusive, on choisit ses formulations avec un souci permanent de lisibilité. Elle doit être pensée comme un outil pédagogique qui s'adresse à tout le monde. Il est intéressant de constater que certains arguments qui lui sont opposés étaient déjà invoqués contre la féminisation des noms de métiers et fonctions. Je pense à l'argument subjectif de l'esthétisme, qui semble méconnaître la part que joue l'habitude dans notre appréhension des mots. Des termes comme « autrice » ou « poétesse » étaient encore d'usage jusqu'au XVII siècle pourquoi ne pas se les réapproprier ? Je pense également à l'argument de la neutralité du masculin, qui repose sur l'idée qu'il y aurait une dualité : d'un côté, un masculin neutre générique ; de l'autre, un masculin spécifique désignant l'homme. Or les psycholinguistes qui se sont penchés sur cette question soulignent que le masculin dit « générique » s'efface toujours devant le masculin « spécifique »- lorsqu'on prononce le mot « sénateur », on se représente en premier lieu un homme. La féminisation des noms de métiers et fonctions a longtemps été vivement décriée ; elle rencontre d'ailleurs toujours des résistances sur certaines travées de notre hémicycle. Appelée des voeux d'Édouard Philippe dans sa circulaire aux administrations de novembre 2017, elle apparaît désormais comme largement consensuelle, ce dont témoigne l'évolution récente de la position de l'Académie française sur le sujet. sera peut-être l'avenir d'autres techniques d'écriture égalitaire- l'histoire en jugera. Je souhaiterais préciser qu'il n'a jamais été question, ni pour moi ni pour la plupart de celles et ceux qui la défendent, d'obliger de recourir à l'écriture inclusive. Il ne s'agit pas de l'imposer, mais simplement de garantir la liberté de s'en emparer., emparer., celles et ceux qui souhaitent l'interdire s'inscrivent dans une démarche coercitive rigide, se heurtant parfois à la réalité des usages. Tout par une citation d'Éliane Viennot, professeuse émérite de littérature, dont la réflexion sur ces sujets est bien connue : « Réfléchir aux meilleures pratiques de l'écriture inclusive et aux moyens de la diffuser, mesurer sérieusement ses effets psychosociaux et son impact sur les inégalités, n'est-ce pas un programme plus utile que de la peindre, encore et encore, en péril mortel ? La langue est le ciment de notre culture. Réjouissons-nous de la voir pensée, discutée, négociée.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, « la langue française est une femme. Et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, touchante, voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu'on l'aime de toute son âme, et qu'on n'est jamais tenté de lui être infidèle », écrivait Anatole France. Existe-t-il une langue, mes chers collègues, qui incarne mieux le respect de la féminité, le romantisme et la poésie que le français ? Cette langue magnifique, aussi présente dans la littérature que dans la diplomatie, est l'une des racines les plus profondes de notre civilisation et de notre culture. Être Français, c'est d'abord parler français, comme nous le rappelle l'article 2 de notre Constitution. C'est notamment ce qui faisait dire à Albert Camus : « Ma patrie, c'est la langue française. » Aujourd'hui, fini les grands esprits et place aux idéologues et à la déconstruction de ce que nous sommes. Emmanuel Macron veut déconstruire notre histoire ; dans le même élan, on cherche à déconstruire la langue qui fait notre socle commun, qui protège le coeur de notre nation et relie, à travers la francophonie, ceux qui l'aiment et ceux qui s'y retrouvent. Mme de La Fayette, la comtesse de Ségur et George Sand n'étaient pas au courant qu'elles utilisaient une langue sexiste. De cette idiotie est née- et maintenant prospère -l'écriture inclusive, qui n'est rien d'autre qu'une écriture de l'exclusion. En prétendant combattre les inégalités, cette nouvelle dérive met la langue française en grand péril et crée de nouvelles disparités : par la succession des points et des ruptures de mots, les malvoyants, les dyslexiques et les étudiants étrangers sont les premières victimes de ces saccades qui sont autant de saccages. L'abolition du genre, l'obsession sexiste et l'apparition du neutre sont les fossoyeurs du français, alors que le niveau en orthographe des écoliers est déjà affligeant.

Ces militants « linguicides » sont les mêmes qui refusent de commémorer le bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon I, les mêmes qui travestissent la réalité de notre histoire pour imposer aux Français le poison de la repentance perpétuelle, les mêmes qui veulent faire table rase du passé, de notre identité pour nous priver du futur commun. Tous sont porteurs de la même motivation, du même virus mortel : la haine de la France. Leur volonté de la combattre, de l'abattre, passe aussi par la destruction de sa langue,

Inutile de torturer davantage cette oeuvre, ces quelques mots ainsi défigurés suffisent à démontrer toute l'absurdité et le danger que représente l'écriture inclusive pour la beauté et la compréhension de dame ou damoiselle langue française.

les difficultés supplémentaires introduites par l'écriture inclusive dans l'apprentissage et l'appropriation de la langue française, à l'écrit comme à l'oral, auraient dû, à elles seules, clore le débat. En effet, pour les personnes « dys »- dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques -et pour les non-voyants et les malvoyants, elle est sans aucune ambiguïté facteur d'exclusion. La place des femmes dans la société constitue certes un défi éducatif, mais qui ne qui ne saurait occulter l'autre défi majeur que représente l'apprentissage de la lecture chez les jeunes enfants. Ce n'est pas faire injure aux immenses, mais inégales, capacités d'apprentissage des enfants que de reconnaître que la déconnexion entre la logique de la langue écrite et celle de l'oral rendra son appropriation moins fluide. De ce point de vue, et forte de mon expérience d'enseignante, je dois dire d'emblée que j'approuve la ferme position du ministre de l'éducation en faveur de l'interdiction de l'écriture inclusive dans l'enseignement. De fait, si une langue a vocation à évoluer avec la société, sa structure ne devrait ni se déconstruire ni se dénaturer pour s'enrichir. Par surcroît, jusqu'ici, la langue française a plutôt suivi un mouvement naturel, et inclusif, de simplification.

au point médian vient détourner l'usage de ce signe de ponctuation qui indique la fin d'une phrase selon la règle « une phrase commence par une majuscule et se termine par un point » et qui sert la compréhension des textes. En détournant la ponctuation, l'écriture inclusive ne féminise pas seulement les mots, elle modifie les structures grammaticales et orthographiques de l'écriture. J'observe d'ailleurs que l'effet dominateur des hommes sur les femmes, lequel résulterait de la règle selon laquelle

fait revenir au point de départ ! Pourquoi, dès lors, ne pas faire évoluer la formulation de la règle ? Si l'on veut transformer les mentalités avec l'écriture, ce même objectif peut être atteint par l'enseignement de la distinction entre entre le genre des mots et le sexe des personnes, moins complexe et permettant d'éviter l'assignation au sexe de la personne. De fait, un autre grand risque de l'écriture inclusive est à mon sens celui de l'essentialisation des femmes. Dans cette logique, la facteure, l'autrice, les défenseures, les actrices sont distinguées d'abord en tant que femmes, ce qui conduirait à terme au même effet pour les hommes. Mais à l'heure où notre époque refuse les déterminismes de genre, afin de permettre aux transgenres ou encore aux personnes qui ne souhaitent pas être déterminées de trouver pleinement leur place, il me semble qu'une reconfiguration de l'écriture à partir d'un axe binaire masculin/féminin irait à rebours de la société. Visuellement, le point n'inclut pas, mais établit une séparation entre la forme masculine et la marque du féminin. De nombreux linguistes ont démontré le caractère en réalité « excluant excluant » de ce mode d'écriture, qui déplace un sujet sociétal sur le terrain de la grammaire. Trente-deux d'entre eux ont ainsi publié une tribune collective pointant « outre les défauts fonctionnels » de l'écriture inclusive, l'absence de lien linguistique exclusif exclusif entre la féminisation des mots et la féminisation de la société et confirmant, en tout état de cause, l'effet d'éviction pour les personnes présentant des difficultés d'apprentissage.

par une agence de communication, qui conduit à établir une distinction entre genre des mots et sexe des personnes. Ce sont donc toutes ces raisons qui conduisent à considérer que l'écriture inclusive exclut plus qu'elle n'inclut. Dans cette optique, notre attention doit être concentrée sur les enfants. Nous devons nous garder de leur ajouter une contrainte supplémentaire, alors que les positions de la France au classement PISA nous éclairent sur les enseignements à conforter. La féminisation des mots ou l'écriture épicène, qui privilégient les genres neutres, sont des vecteurs de visibilité pour les femmes, laissant à chacun le choix de les utiliser selon son appréhension de la langue. Le français est suffisamment riche

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, avant d'entamer mon propos, je tiens à saluer le travail remarquable de ma collègue Annick Billon en tant que présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes. La reconnaissance des droits des femmes est un sujet universel, qui ne doit pas seulement être porté par les femmes. Ce combat nous concerne tous et doit aussi être mené dans la langue française. Par exemple, les titres et les fonctions se féminisent, car de plus en plus de femmes occupent des postes qui étaient autrefois détenus par les hommes. La langue n'est pas figée et s'adapte à l'évolution de la société. Cependant, l'évolution de la visibilité des femmes ne doit pas se faire au prix d'une dénaturation de la langue. L'écriture inclusive est à ce titre une aberration. Les défenseurs de l'écriture inclusive se fondent sur la règle du « masculin l'emporte sur le féminin » pour prouver que les femmes ont été exclues de la langue française. Or il ne s'agit ici que d'un masculin grammatical. Personne ne peut voir dans cette règle la transposition d'une supposée prédominance de l'homme sur la femme, comme ils voudraient nous le faire croire. Il faut arrêter de voir dans la langue française la retranscription d'une société patriarcale où le mâle dominant l'emporterait sur la femelle dominée. Si nous n'écrivons plus comme au XVI siècle, à la manière du poète Ronsard, « la rose qui ce matin avait déclose », c'est parce que le peuple, dans sa sagesse, a fait prévaloir le masculin, à la manière d'un genre neutre, car le féminin était trop difficile à prononcer. L'écriture inclusive constitue une atteinte à la mémoire collective et à la construction de notre langue, qui a été façonnée par le peuple français au fil des siècles. Ceux qui croient que notre langue est misogyne parce qu'elle serait « genrée » oublient que c'est la marque des langues latines comme l'italien ou l'espagnol. D'ailleurs, les genres ne sont qu'arbitraires : les un zèbre » ou « un éléphant » désignent aussi bien le mâle que la femelle. Si le français exclut le féminin, comment expliquer que notre langue ait féminisé les piliers de notre société : la liberté, la démocratie, la République, la fraternité ? Il y en aurait tant d'autres à citer Les hommes devraient-ils à leur tour s'émouvoir et se sentir exclus lorsque les mots qui les caractérisent ont un genre féminin ? Un homme peut très bien être « une sentinelle », « une sage-femme » ou « une nouvelle recrue Cette écriture inclusive n'est pas seulement illisible et imprononçable ; elle est aussi un « péril mortel » aux yeux de l'Académie française. Dans la mesure où le parler sera différent de l'écrit, il n'y aura plus d'unité, car l'écriture ne retranscrira plus le langage. Cette déconstruction par pure idéologie entraîne également de nombreuses difficultés pour l'apprentissage. Quand on sait que 25 % des élèves qui arrivent en sixième ont des difficultés pour lire et écrire, on se demande pourquoi il faudrait ajouter de la complexité à l'une des langues les plus difficiles au monde. la députée Clémentine Autain écrivait le 29 mai 2018 sur Twitter : « Nous refusons que les droits de nos enfants, étudiant.e.s, élèves, soient à ce point bafoué.e.s. » « Bafoué » se rapporte ici à « droits » : c'est donc une erreur que de l'écrire au féminin. Si même les chantres de l'écriture inclusive se mettent à faire des fautes, comment voulez-vous que nos enfants s'y retrouvent ? Pensons également à nos amis francophones ! Si les pays du Maghreb, d'Afrique ou le Canada rejetaient l'écriture inclusive, il y aurait alors une rupture de la francophonie. Notre langue s'en trouverait désunie et de moins en moins parlée dans le monde. Il y a donc une différence fondamentale entre une évolution imposée par l'idéologie politique et une évolution naturelle tenant compte des mutations de la société. En 2021, près de 150 mots sont entrés dans le dictionnaire, comme « black bloc », « dégagisme » ou « féminicide ». Greta Thunberg a même fait son entrée dans la catégorie des noms propres ! Ces mêmes idéologues nous expliquent depuis des années que le sexe ne doit pas être assimilé à l'identité de genre. Et voilà que, à propos de l'écriture, ils considèrent que le genre grammatical est le reflet de leur vision de la société, où la femme serait dominée par l'homme. Pour terminer, je reprendrai un extrait de la tribune écrite par trente-deux linguistes dans le journal en septembre 2020 En introduisant la spécification du sexe, on consacre une dissociation, ce qui est le contraire de l'inclusion. En prétendant annuler l'opposition de genre, on ne fait que la systématiser. » L'écriture supposément « inclusive » entraîne, en réalité, une exclusion réciproque entre les hommes et les femmes. La parole

Le langage inclusif, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord la féminisation des noms de métiers, de fonctions et de personnes. L'écriture inclusive ne concerne jamais ni les choses ni les concepts. Par exemple,

les femmes ne se reconnaissent pas quand on parle de « droits de l'homme ». Je pourrais éventuellement suivre ceux qui me disent que les droits de l'homme concernent aussi les femmes. Ce serait vrai si les droits de l'homme avaient concerné les femmes.

soit. Sur quoi porte le désaccord ? D'abord, peut-être, sur notre constat de l'effet du masculin générique. Je pense que le masculin générique, et des linguistes le pensent avec moi, excluent les femmes. Il ne permet pas de représenter et de visibiliser les femmes. les femmes. Nous travaillons les uns et les autres à permettre une meilleure visibilité des femmes dans la langue. Nous avons les mots épicènes, qui ont été évoqués. Nous avons aussi le point médian.

ce débat aujourd'hui, il y a une circulaire du Premier ministre et une déclaration du ministre de l'éducation nationale ... Ce n'est pas sérieux ! La bataille contre le point médian est devenue une bataille politique. C'est une bataille de résistance à l'évolution de la société.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, si les langues ont vocation à permettre aux hommes de communiquer entre eux, il est permis de convenir que le français a poussé assez loin cette logique, jusqu'à l'universel. Après avoir été la langue de la diplomatie européenne, il a été celle de l'olympisme, et la France détient toujours le record du nombre de prix Nobel de littérature. En cela, c'est un bien collectif. Aucune faction ne devrait pouvoir le confisquer pour servir ses intérêts. Le français est une langue syllabique, qui implique de pouvoir lire à haute voix sa forme écrite. C'est aussi une langue irrégulière, dont l'apprentissage est réputé difficile. Malgré cela, nous observons que certains militants s'activent pour la complexifier en ajoutant un nouveau mode grammatical : l'inclusif. Ils la parasitent de déclinaisons imprononçables et de pronoms fantaisistes, non pas pour la nourrir, puisque, après tout, la langue est un organe vivant, mais pour la refonder et substituer au français un idiome seulement compréhensible d'un groupe de locuteurs, qui, sous le masque de l'égalité, cultive l'entre-soi d'une avant-garde éclairée. Un tel sabir visant à se démarquer pourrait nous divertir, comme le faisaient les vieux jargons français d'autrefois, tels le javanais, le louchébème ou même le verlan, qui remonte au XII siècle. Sauf qu'aujourd'hui les facéties des promoteurs de l'écriture dite inclusive ne nous amusent plus : nous sommes passés de Queneau à Orwell, de l'argot à la novlangue Du camp de ses partisans, j'entends monter le contentement de renverser les statues de linguistes distingués disparus il y a trois ou quatre siècles. Ce ne sont pas eux qu'ils touchent. En imposant leurs écrits indéchiffrables, ils sapent en réalité le patient travail de nos instituteurs et de nos professeurs de français, qui s'efforcent de transmettre à leurs élèves, dont le français n'est parfois pas la langue maternelle, l'autonomie dans la lecture et l'écriture, donc dans la vie. Malgré cela, en fin de troisième, 15 % des collégiens ne maîtrisent pas le français ou le maîtrisent mal. En outre, 27 % des entreprises ou administrations interrogées déplorent régulièrement des problèmes causés par l'incompréhension de la langue écrite. Les orthophonistes nous alertent sur les difficultés bien réelles engendrées par l'inclusif pour la lecture des dyslexiques, sans parler de celles qui sont rencontrées par les malvoyants et les personnes âgées. Alors, c'est vrai, en français, le genre neutre est porté par le masculin. Cette règle date du XVII siècle, époque à laquelle l'Académie a voulu encadrer l'usage d'une langue encore adolescente. Mais est-ce vraiment la grammaire qui a mis les femmes en état de minorité ? Lui faire porter cette responsabilité au nom de la « représentation mentale » induite ne me semble guère étayé., le persan, le chinois ou le turc ne distinguent pas les genres : sont-ils pour autant des facteurs de libération pour leurs locutrices ? Cependant, et par définition, une langue vivante n'est pas inerte. Je me réjouis en cela de la féminisation des métiers et des fonctions qui ont tant tardé à être exercés par des femmes. Mais n'embrigadons pas notre langue ! N'en faisons pas un ferment de division, alors qu'elle doit rester ce terrain d'entente et, donc, de dialogue. Miner la structure même de la langue, c'est signifier aux individus d'une société qu'ils n'ont plus d'essence commune, qu'ils n'ont plus vocation à s'adresser les uns aux autres, finalement plus rien à faire ensemble. Or, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, aujourd'hui, notre société a davantage besoin de traits d'union que de points médians. La parole est

Voilà, madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis heureuse, après vous avoir attentivement écoutés, de m'exprimer au nom du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la question de l'écriture inclusive. Si le sujet est aujourd'hui débattu dans cet hémicycle, c'est bien, et cela a été rappelé à plusieurs reprises, parce que nous ne parlons pas d'un petit sujet, d'une lubie de quelques personnes isolées qui se seraient prises de passion pour un nouveau jeu littéraire. L'écriture inclusive n'a rien à voir avec un exercice de style. Elle est un enjeu de société, un enjeu à la fois éducatif et politique, c'est-à-dire un enjeu qui nous préoccupe tous. Que l'on ne s'y trompe pas. Je ne parle pas ici de l'évolution nécessaire de la langue et des usages consistant à accorder les métiers et les fonctions selon le genre. Cette évolution est un progrès évident, que nous saluons, salutaire pour les femmes et pour la société dans son ensemble. Je ne parle pas de la féminisation des noms, mais bien de l'écriture dite « inclusive », au sens où l'entend la circulaire du Premier ministre Édouard Philippe du 21 novembre 2017, à savoir en tant que « pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l'emploi du masculin, lorsqu'il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l'existence d'une forme féminine ». En clair, nous parlons bien aujourd'hui du point médian et des néologismes dits neutres, comme le pronom non binaire « iel », censé remplacer à la fois le « il » et le « elle ». Cette écriture dite « inclusive » prend de l'essor et dépasse aujourd'hui très largement la sphère militante ou associative. On la retrouve désormais dans certains journaux, on la voit exploser sur les réseaux sociaux, on ne s'en étonne plus dans la communication des entreprises ni dans les publicités de marques grand public. Nul n'ignore aussi combien son usage s'est répandu à l'université, dans certains intitulés de cours, de travaux dirigés ou de publications. Certains professeurs, que je crois volontiers peu nombreux, approuvent de telles pratiques et l'encouragent même, au détriment d'élèves ou d'étudiants qui ne voudraient ou, tout du moins, ne sauraient en faire usage. De même, à l'université, et désormais à l'école, de plus en plus d'élèves l'emploient dans leurs copies, et nos professeurs se trouvent bien en peine

qui prétend lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes et manifester la diversité du genre humain ? Pourquoi prendre le risque de se mettre à dos un, sinon plusieurs, élève ou collègue ? Comment ne pas plier face aux pressions, aux intimidations parfois, car elles existent, sommant d'y avoir recours ? Face à cela, il est une réponse : l'institution. L'institution, c'est-à-dire l'État, doit se prononcer avec clarté et fermeté sur un tel sujet, car elle est la seule à pouvoir fixer la norme à laquelle chacun peut se référer en toutes circonstances. Quatre ans après la circulaire de 2017 et l'avertissement de l'Académie française, je veux donc le redire avec la force et avec la conviction que seule donne l'évidence : l'écriture inclusive est un danger pour notre école

Je commencerai par parler de l'école. L'écriture dite « inclusive » vient battre en brèche la mission première de tout système éducatif apprendre à lire. Nul ne peut contester les difficultés de lecture qu'entraîne déjà pour l'adulte une telle graphie. L'écriture inclusive nous fait buter sur les mots, nous contraint au bégaiement. Elle rend la marche d'un texte chaotique, elle disloque les mots en les fendant en deux. L'écriture inclusive nous contraint à la myopie : on ne voit plus que le mot écrit, on ne voit pas plus loin que le mot, on oublie le sens de la phrase, finalement le sens tout court. L'écriture inclusive marque le retour au stade du déchiffrage ; elle est une régression de l'acte de lire. Chacun peut donc imaginer combien ces difficultés de lecture sont décuplées chez le jeune enfant qui apprend à lire. Vous le savez sans doute, madame la sénatrice, en classe de CP, les élèves apprennent à associer les lettres, dont la combinaison produit des sons, qui se combinent en mots. Ces mots font ensuite des phrases, dont l'enfant comprend enfin le sens. Il ne faut pas moins que l'association de cinq étapes successives pour apprendre à lire. Tous les enfants ont besoin de règles claires. Aucun élève n'apprend dans le flou. Pour l'apprentissage de la langue française, les programmes scolaires se réfèrent aux normes orthographiques et grammaticales en usage, et les mêmes règles sont enseignées à tous. La clarté de la norme est la condition indispensable de la transmission. À l'opposé exact de cela, les militants de l'écriture inclusive font évoluer leurs propres règles syntaxiques au gré des semaines. On ne compte plus les querelles intestines pour décider à quel endroit exactement placer le point médian, quels accords privilégier, jusqu'où aller dans le démembrement de la phrase. L'écriture inclusive a ses radicaux et ses modérés,

En dépit d'un progrès indubitable depuis 2018, à l'entrée en sixième, un nombre encore trop important d'élèves présente des difficultés de déchiffrage manifestes, qui sont inquiétantes. De fait, l'écriture inclusive constitue bien un obstacle pour l'acquisition de la langue et de la lecture pour la très grande majorité des enfants, sinon pour tous. Comme l'a écrit récemment le professeur émérite Bernard Cerquiglini, l'écriture inclusive rompt avec le courant progressiste, qui, depuis le XVI siècle, milite en faveur d'une lisibilité démocratique de l'écrit. Il est donc tout à fait exact de parler d'écriture excluante. L'écriture inclusive est excluante au moins à un autre titre : elle est inadaptée aux élèves présentant des troubles d'apprentissage. Je pense en particulier aux enfants atteints de dyslexie, de dyspraxie ou de dysphasie. Je pense aussi à tous les enfants en situation de handicap, enfants autistes, enfants malvoyants, qui dépendent de logiciels d'aide à la lecture incapables de reconnaître l'écriture inclusive et, donc, de restituer le texte lu. Aussi, la typographie de l'écriture inclusive- une typographie qui ne se lit pas et ne se dit pas, une typographie instable, qui dépend du bon vouloir créatif de chacun, une typographie incapable de se choisir une règle orthographique plutôt qu'une autre -n'a en vérité -n'a en vérité aucunement sa place dans notre école. Et aucun avenir ! Par conséquent, parce que nous défendons une école véritablement inclusive,

le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports vient de publier une circulaire proscrivant son usage dans les enseignements. Très bien ! Elle viendra conforter nos élèves dans leurs apprentissages et conforter nos professeurs dans leur travail. Mesdames, messieurs les sénateurs ? S'il vous plaît ! ... nous pourrions nous en tenir à souligner l'inadéquation fondamentale entre écriture inclusive et apprentissage de la lecture. Caricature ! Autrement dit, nous pourrions nous en tenir à l'école. L'école est le creuset de la République. L'école a tout à voir avec la République, et ce qui touche aux principes fondamentaux de notre République touche nécessairement à notre école. Beaucoup a déjà été dit cet après-midi sur les dangers que constitue l'usage de l'écriture inclusive pour notre langue et pour notre pays. Vous avez ainsi parlé de la francophonie. comme s'en est inquiétée l'Académie française, je suis convaincue que la généralisation de l'écriture inclusive, qui complexifie abusivement notre grammaire et notre orthographe, qui ne sont déjà pas si simples, marquerait la mort annoncée de la pratique de la langue française dans le monde. Rappelons qu'il n'y a pas d'accord des adjectifs en anglais et quasiment pas d'accord des verbes non plus. Cette simplicité est un avantage compétitif évident pour la diffusion de l'anglais dans le monde. Tout autre est le cas des langues romanes, qui nécessitent connaissance du masculin et du féminin de chaque nom et accord des adjectifs. Dans cet environnement linguistique déjà complexe, les tenants de l'écriture inclusive, en refusant d'accorder au masculin sa fonction de neutre, font le choix assumé d'accroître considérablement les difficultés préexistantes de notre langue par l'excroissance artificielle des mots. Par conséquent, avec l'expansion de l'écriture inclusive, la langue anglaise, déjà en situation quasiment hégémonique à travers le monde, gagnerait à coup sûr et probablement définitivement sur la langue française. Je parle de l'anglais, mais je pourrais parler de bien d'autres langues.

« L'histoire de France commence avec sa langue », nous dit Michelet. Nous sommes les dépositaires temporaires des mots, des voix, des âmes qui ont sculpté la langue française par le passé. Par nos vies, nous sommes les bâtisseurs de la langue que, à notre tour, nous devons transmettre.

Cette vérité appelle l'humilité et doit tempérer l'hubris de quelques-uns. Cette vérité doit aussi nous pousser à réfléchir par deux fois avant d'accepter des évolutions moins dictées par l'usage courant que par la nouvelle doxa du temps présent. Cela a été dit, l'écriture inclusive participe d'une idéologie qui, comme toute idéologie, ne souffre pas la contestation et dont les partisans cherchent au contraire à imposer leurs vues à tous. Cette idéologie oppose les hommes et les femmes, les dominants et les dominés. Elle fait du terrain linguistique un champ de bataille où deux camps combattent face à face. Sans doute vaudrait-il mieux éviter dans un cours de grammaire de dire que « le masculin l'emporte sur le féminin ». En revanche, on peut tout simplement dire qu'au pluriel le mot s'accorde au masculin, qui, dans la langue française, fait office de neutre. L'écriture inclusive est donc le refus du neutre, c'est-à-dire de l'universel. L'écriture inclusive, c'est rendre visible le genre et rendre invisible l'universel. Ce mouvement d'inversion de la norme est en contradiction totale avec les principes mêmes de notre République, qui rassemble avant d'exclure, qui unit avant de séparer. Par conséquent, l'écriture inclusive n'est pas seulement illisible, inintelligible, impraticable et préjudiciable aux apprentissages, pas uniquement le choix délibéré d'exclure une partie de nos concitoyens, ! ... elle est une méconnaissance absolue et, je crois, voulue de notre langue et de son histoire, une tentative d'appauvrissement de notre manière de penser et, plus encore, de nous penser. Mesdames, messieurs les sénateurs, l'école de la République apprend à chaque élève à habiter sa langue, c'est-à-dire à être porté par une littérature qui a toujours célébré cet esprit de liberté et de partage qu'est l'esprit français. Notre langue est davantage qu'un trésor : elle est notre destinée commune. C'est par la langue que nous devenons nous-mêmes et que nous nous projetons au-delà, vers cet universel qui caractérise le rapport si singulier que les Français entretiennent avec le monde.

l'heure était venue de déposer une proposition de résolution en faveur de l'association de Taïwan aux travaux de plusieurs organisations internationales.

Nous sommes dans une situation marquée par la séparation de Taïwan et de la Chine continentale depuis 1949, à l'issue d'une guerre civile de plus de vingt ans qui s'est conclue par la prise de pouvoir du parti communiste chinois et l'instauration de la République populaire. La France, puis les États-Unis et, à leur suite, la plupart des États de la communauté internationale ont reconnu le régime de Beijing comme le représentant de toute la Chine.

et, d'autre part, une société de plus en plus libre et ouverte, avec des élections réellement libres et pluralistes, une presse libre, un développement scientifique et culturel débarrassé des censures. Du côté de la Chine continentale, nous savons que l'évolution est différente. Les autorités de la Chine populaire ont toujours affirmé leur volonté de faire revenir Taïwan dans leur souveraineté. À cette fin, elles ont formulé dès les années 1980 la doctrine « un pays, deux systèmes », qui, on le sait, a été appliquée ensuite à Hong Kong, avec l'évolution ultérieure que nous observons. À des périodes diverses, ces autorités ont exercé des pressions militaires à proximité de Taïwan, soutenues par des lois prévoyant l'emploi de la force au cas où Taïwan déclarerait formellement son indépendance. Ces pressions militaires se sont renforcées au cours des deux dernières années en cohérence avec la montée très prononcée des capacités de défense de la Chine populaire. La France conduit toute son action internationale dans le cadre du multilatéralisme organisé et, donc, des institutions internationales où les États prennent ensemble des mesures de régulation ou de promotion destinées à améliorer le sort des citoyens du monde, au sein duquel priment leur sécurité et leur santé. pays souhaite logiquement qu'une entité comme Taïwan, dont la contribution à la vie internationale est importante dans de nombreux domaines, puisse y être entendue.

Il est évident que c'est le cas de Taïwan dans bien des champs d'action, le plus emblématique étant bien sûr celui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), compte tenu de l'expérience éclatante de l'île en ce qui concerne la gestion de la pandémie mondiale

à notre exécutif pour qu'il continue ses interventions en partage avec d'autres puissances. Le point saillant relevé dans notre texte est que les autorités de la République populaire de Chine ont accepté que Taïwan participe aux travaux de l'OMS pendant plusieurs années,

qu'elle entendait respecter le entre les deux rives du détroit, ce qui se confirme dans les faits depuis cinq ans. Nous sommes donc fondés à estimer respectueusement que la République populaire de Chine pourrait, sans infléchir ses positions de fond, accepter à nouveau une collaboration des représentants de Taipei à l'Assemblée annuelle de l'OMS et, par conséquent, aux outils concrets de coopération en faveur de la santé mondiale qui y sont discutés. En sollicitant de tous nos collègues un soutien à cette proposition de résolution dont l'inspiration est constructive et conciliatrice, nous entendons- je veux le dire très clairement -respecter la loi internationale ... Il faut conclure,

En cohérence avec la conduite constante de la France sur cette question, nous ne pouvons que recommander la retenue et la recherche de solutions pacifiques et négociées. La proposition de résolution soumise à votre approbation, mes chers collègues, s'inscrit sans équivoque dans cette ligne. Nous vous la soumettons par conséquent

pour tous dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé, à lutter contre la criminalité transnationale Interpol, à assurer la sécurité aérienne civile internationale sous l'égide de l'Organisation de l'aviation civile internationale et, enfin, à trouver des solutions viables pour le changement climatique climatique grâce à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Tous ces sujets impliquent nécessairement des efforts concertés de la part de toutes les nations et la participation de tous les citoyens du monde vivant sur notre planète. Les différences d'opinions politiques doivent être mises de côté, car ces questions essentielles dépassent les frontières. S'agissant de la santé, cet état d'esprit est d'ailleurs bien retranscrit dans la Constitution de l'OMS : « La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. » Pourtant, Taïwan ne peut pas participer aux travaux de l'OMS ni à ceux des autres instances internationales spécialisées, ce qui ne se justifie pas. La superficie de Taïwan est proche de celle des Pays-Bas et sa population équivalente à celle de l'Australie. L'île a un PNB légèrement supérieur à celui de la Suède ou de la Turquie. Taïwan importe plus que la Russie, l'Australie ou le Brésil et exporte davantage que l'Espagne ou l'Inde. Les relations commerciales de Taïwan un niveau proche de celles de la Norvège, et, si l'on considère le volume d'échanges avec la France, ce pays est un partenaire plus important pour nous que la Thaïlande, le Nigéria, la Malaisie, l'Indonésie ou l'Australie. La France a des intérêts dans cette partie du monde. Taïwan produit 84 % des semi-conducteurs les plus sophistiqués utilisés sur la planète. Comme vous le savez, mes chers collègues, notre industrie automobile en dépend. En raison de l'importance des échanges internationaux que ces activités économiques engendrent, il est anormal que Taïwan, qui dispose de deux compagnies aériennes réputées mondialement, ne puisse pas participer aux débats concernant la sûreté aérienne, les services de navigation, la protection de l'environnement et les questions économiques. De même, avec l'augmentation constante des passagers qui transitent par Taïwan, il est regrettable que ce pays soit exclu d'Interpol, alors que nous souhaitons accentuer nos efforts pour lutter contre le terrorisme, le trafic de drogue et toutes les formes de criminalité. S'appuyant sur des valeurs démocratiques profondément ancrées, Taïwan a été largement saluée à travers le monde pour son excellente gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19. À ce jour, on dénombre un petit millier de personnes infectées et on déplore seulement une dizaine de décès. Il convient de souligner que Taïwan a offert 54 millions de masques chirurgicaux et des fournitures destinées à contrer la pandémie à plus de 80 pays. En effet, ce pays partage avec la France un attachement fondamental à la démocratie et aux valeurs universelles. Les principes démocratiques qui prévalent à Taïwan sont une source d'inspiration. À Taïwan, toute personne peut librement s'exprimer, et les journalistes ne connaissent pas pas la censure. Taïwan est considérée comme le pays le plus libre d'Asie, au même niveau que la France. Les femmes ont un statut égal à celui des hommes. Non seulement c'est une femme qui a été élue à la présidence et qui dirige le pays depuis cinq ans, mais 42 % des sièges à l'Assemblée nationale taïwanaise Taïwan est tout à fait à même d'apporter une contribution efficace dans les domaines que j'ai évoqués. Encore faut-il laisser ce pays occuper la place qui lui revient dans les instances internationales. Malgré la prospérité et la stabilité de cet État, le célèbre hebdomadaire britannique vient d'illustrer sa couverture du 1 mai 2021 en soulignant que Taïwan était l'endroit le plus dangereux de la planète en raison de la menace militaire de la Chine qui pèse sur l'île La paix et la prospérité de cette région sont importantes pour l'ensemble du monde. Nous devons travailler ensemble à les préserver. La question du bien-être de l'humanité est au coeur de nos préoccupations. C'est tout le sens de notre démarche aujourd'hui. André Malraux a dit à propos de l'établissement des relations diplomatiques avec la Chine populaire : « Marchons ensemble, mais sans mélanger nos drapeaux ! » Alors, oui, marchons, travaillons, coopérons avec la Chine, mais sans nous écarter de nos valeurs essentielles et en respectant chaque drapeau. Il convient de tous les inclure, celui de Taïwan compris, car il s'agit d'une question majeure qui concerne notre avenir commun. La

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens à remercier nos collègues Alain Richard et Joël Guerriau de nous permettre de débattre de la situation de Taïwan. Depuis que les forces communistes chinoises ont remporté la guerre civile et pris le contrôle du continent en 1949, ce pays essaie de préserver son autonomie. Le développement économique de ce territoire a été et reste particulièrement remarquable. Avec un PIB comparable à celui de la Suisse ou de la Suède, Taïwan fait partie des premières puissances économiques asiatiques. Taipei est en outre un acteur incontournable de la production mondiale des semi-conducteurs les plus avancés. Ces puces sont nécessaires aussi bien à l'industrie automobile qu'à celle du numérique ou à celle de l'armement. Ses entreprises conservent, dans ce domaine, une avance de près d'une décennie sur leurs concurrents. Le miracle taïwanais a fait de l'île l'un des quatre dragons asiatiques et a permis à la population de bénéficier d'un niveau de vie équivalent à celui de la population de l'Union européenne. Dans le domaine de la santé, l'île a démontré des compétences indéniables. Elle a fait face avec succès à plusieurs épidémies, dont celle de la covid-19. Alors que Taïwan compte plus de 23 millions d'habitants, le pays a su limiter les contaminations tout en préservant son économie : elle ne déplore ainsi qu'une dizaine de décès

au sein de différentes instances internationales. Cette initiative a été saluée par la Présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, qui a souligné la pertinence de telles coopérations.

que Taïwan puisse faire bénéficier la communauté internationale de ses compétences dans des matières aussi diverses que la santé, la coopération policière, le dérèglement climatique ou encore l'aviation civile. de résolution est également l'occasion de réaffirmer notre attachement aux principes du multilatéralisme, du dialogue et de la coopération au sein de la communauté internationale. Ces principes sont au fondement d'une paix et d'une stabilité durables. Taïwan est en effet l'objet de vives tensions géopolitiques impliquant la Chine et les États-Unis. La région assiste depuis quelque temps à une importante montée en puissance des forces armées, et singulièrement des forces navales. Ce climat de course aux armements laisse craindre l'éclatement d'un conflit ouvert dans les prochaines années. Un tel conflit serait bien entendu tragique pour les acteurs de la région. néfastes de celui-ci s'étendraient certainement à l'ensemble de la communauté internationale. Nous sommes convaincus que la paix et la coopération ont fortement contribué à la prospérité des pays de la zone. Il nous semble qu'il est donc dans l'intérêt de tous de veiller à les préserver. Cette voie constitue également la suite logique des relations pacifiques qui prédominent jusqu'à présent et qu'il importe de perpétuer. Dans la mesure où cette proposition de résolution ne comporte aucune reconnaissance de l'indépendance de Taïwan, elle ne constitue pas une remise en cause de la position française.

Renforcer l'intégration de Taïwan dans les instances internationales permettra de faire profiter de précieuses synergies. C'est aussi l'occasion d'éloigner un peu plus la perspective d'un conflit qui ne profiterait à personne. Le dialogue et la coopération fourniront des réponses durables aux nombreuses tensions qui pèsent sur cette région. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants espère que ce texte recevra un large soutien de notre assemblée. La parole

Depuis 2016, elle ne dispose plus de sa place d'observateur à l'Assemblée mondiale de la santé, en conséquence de quoi elle ne peut plus être associée aux réunions de l'Organisation mondiale de la santé. Rien ne peut légitimer la mise à l'écart d'un système politique dont nous connaissons tous ici les mérites, tant en termes de vie démocratique que de politique sociale et éducative et de protection de l'environnement. Le contexte pandémique actuel jette toutefois une nouvelle lumière sur l'exclusion de Taïwan des différentes instances de la communauté internationale. La gestion de la crise sanitaire par Taïwan est en effet un modèle pour bon nombre de gouvernements à l'échelon mondial. La densité de la population y est exceptionnellement élevée.

Nous considérons que cette attitude coopérative et pacifique, tournée vers le monde, est représentative de la volonté constante de Taïwan de participer aux organisations internationales en matière de santé, mais aussi à l'Organisation de l'aviation civile internationale, à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à Interpol. Il nous semble évident que cette participation, qui est autorisée pour certaines entités non étatiques, serait éminemment profitable aux différentes organisations. Nous nous prononçons donc en faveur de la présente proposition de résolution. Nous comprenons que cette perception est aussi celle qui sous-tend la position française à l'égard de Taïwan, comme l'a rappelé à plusieurs reprises le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Nous sommes donc confiants dans l'accueil qui sera réservé à cette proposition de résolution et dans les démarches que la France poursuivra en ce sens, en amont de la soixante-quatorzième réunion de l'Assemblée mondiale de la santé qui se déroulera à partir du 24 mai. Nous resterons bien entendu vigilants sur ce point.

Le soutien français à l'association de Taïwan aux instances internationales, bien qu'il n'ait pas pour objectif de reconnaître un statut d'État à ce pays ou de remettre en cause le principe d'une seule Chine, ne sera pas sans conséquences sur nos relations avec Pékin,

Alors, pour sauvegarder l'approche multilatérale et les valeurs démocratiques et humaines qui sont au fondement de notre politique étrangère, quel poids devons-nous accorder aux exigences de Pékin ? Aujourd'hui, le refus de transiger sur nos propres exigences n'est plus une proposition idéaliste, mais une nécessité reconnue comme telle par l'Union européenne qui, après de premières sanctions, a annoncé avant-hier la suspension de la ratification de l'accord d'investissement avec la Chine. C'est aussi un devoir pour la France, aux côtés d'une administration Biden qui fait preuve de fermeté à l'égard de la Chine et de la Russie, de replacer les droits humains et les valeurs démocratiques au coeur de son action diplomatique. Après une présidence Trump tendue et conflictuelle, la responsabilité de notre pays est de s'associer à cette entreprise de reconstruction d'une culture démocratique internationale. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires soutiendra cette proposition de

Située à quelque cent trente kilomètres des côtes chinoises, l'île de Taïwan est un carrefour stratégique qui entretient, depuis plusieurs siècles, des liens d'importance avec l'Europe et la France.

C'est d'ailleurs sur l'initiative de ce groupe que la proposition de résolution à l'étude aujourd'hui a été déposée par vingt-deux de nos collègues, issus de la plupart des familles politiques. Au printemps de l'an passé, lors du confinement strict qu'a connu notre pays, nous étions déjà cinquante et un sénateurs à signer un appel international demandant à l'Organisation mondiale de la santé de la santé de collaborer pleinement avec Taïwan, une manière de reconnaître l'exceptionnelle maîtrise dont ce territoire a fait preuve face à la pandémie de covid-19. En un an et demi, cette île peuplée de plus de 23 millions d'habitants n'a en effet enregistré qu'une dizaine de décès liés à ce terrible virus, un exploit obtenu grâce à des mesures sanitaires rigoureuses et une expertise hors pair. Durement affectée par la crise du SRAS en 2003, Taïwan était certainement le pays le mieux préparé pour affronter cette nouvelle pandémie. C'est en des termes parfaitement respectueux des équilibres diplomatiques que cette proposition de résolution vise à accorder à Taïwan un statut d'observateur au sein de l'Assemblée mondiale de la santé qui se tiendra prochainement. il n'y a là rien qui déroge au règlement de l'OMS, puisque Taïwan jouissait déjà d'un tel statut avant 2016. Nous sommes persuadés que la communauté internationale ne peut que tirer avantage d'une telle efficience, car l'excellence sanitaire de Taïwan ne concerne pas seulement la lutte contre le covid-19, tant s'en faut. Pour la troisième année consécutive, Taïwan occupe le premier rang mondial selon l'indice des soins de santé publié par le site numbeo.com. De nombreux pays, dont la France, ainsi que 1 700 parlementaires de plus de 80 pays se sont déjà exprimés en faveur d'une telle coopération avec les autorités de Taïwan.

Or, parce qu'on lui refuse tout accès en temps réel aux informations globales et aux actualisations régulières de l'OACI, Taïwan met plus de temps que les autres pour se conformer aux standards et aux recommandations de l'Organisation.

pays membres, soit la quasi-totalité des États de la planète, et qui vise à prévenir et à combattre la criminalité grâce à une coopération policière renforcée. Taïwan accueille chaque année un nombre croissant de voyageurs : le pays

est donc un maillon indispensable du système de sécurité globale, tant pour le combat contre la criminalité et la fraude internationales que pour la lutte contre les trafics illicites et la cybercriminalité. Pourtant, Taïwan n'a toujours pas accès au réseau mondial permanent de communication policière d'Interpol ni à ses dix-huit bases de données criminelles. C'est là un trou de taille dans la raquette sécuritaire internationale qu'il est urgent de combler. Enfin, les auteurs du texte suggèrent que Taïwan puisse également participer aux travaux de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Depuis 2015, Taïwan s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Le pays investit beaucoup activement les actions en faveur de la transition écologique, en particulier dans les pays en voie de développement. La participation de Taïwan aux prochaines sessions de la Conférence des parties serait, à n'en pas douter, bénéfique à tous.

internationale au service du bien-être de toutes les populations. C'est la raison pour laquelle l'intégralité des membres du groupe RDPI votera en faveur de ce texte. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nos collègues auteurs de la proposition de résolution souhaiteraient voir relancées les démarches visant à faire participer Taïwan à de nombreuses organisations internationales. Comment ne pas souscrire à cet objectif ? Oui, nous avons besoin de Taïwan à l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS, eu égard à sa gestion exemplaire de la pandémie de covid-19. Oui, nous avons besoin d'intégrer le plus grand nombre possible de pays à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. La lutte contre le réchauffement climatique est un défi mondial qui doit agréger toutes les démarches volontaires. Comme vous le savez, bien que l'île n'ait pas de représentation légale dans le système onusien, elle s'est unilatéralement engagée à respecter les termes du protocole de Kyoto, ainsi que ceux de la COP21, avec une définition d'objectifs très ambitieuse. Il faut le saluer. Ne faudrait-il pas également associer Taïwan à l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, au bénéfice général de la sécurité et du fret ? Elle occupe une position clé dans la région de l'Asie-Pacifique et contrôle un trafic important avec plus de 1 750 000 vols répertoriés en 2018, partis de dix-sept aéroports taïwanais. Enfin, l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, ne doit souffrir d'aucune brèche. Comme souligné dans le texte de nos collègues, associer Taïwan à la lutte contre la criminalité organisée serait profitable à l'ensemble de la communauté internationale, grâce au partage des dix-huit bases de données policières que gère Interpol. D'une façon générale, il est évident qu'il faut rassembler le plus largement au sein des grands outils de coopération internationale. On connaît les vertus du multilatéralisme : il fait progresser de grandes causes comme celles que je viens de décliner. Mais pas seulement ! Il fédère des pays autour d'objectifs communs : c'est aussi construire un monde de dialogue et d'échanges plus propice à la paix que les postures d'isolement. Toutefois, soyons clairs, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, il nous faut trouver un équilibre pour préserver les relations de notre pays avec les deux côtés du détroit de Formose. Nous connaissons l'enjeu géopolitique régissant les relations complexes et passionnelles entre Taïwan et la Chine. Taïwan a un statut particulier. Elle est cependant un interlocuteur fiable pour l'Occident et un acteur économique de premier plan. Je rappellerai juste que son économie est classée au vingt-deuxième rang mondial. Pour la France, Taïwan a représenté un marché à l'exportation de 1,8 milliard d'euros en 2019. Nous lui vendons des biens d'équipement, mais aussi de l'agroalimentaire, bien que Taipei impose à nos viticulteurs de regrettables et lourdes taxes sur le champagne- je tenais à le signaler De l'autre côté, mes chers collègues, il n'est pas besoin de démontrer que la Chine est un partenaire économique incontournable à l'échelle mondiale. Le Gouvernement l'a rappelé ici même en mars dernier. Ce constat invite donc au compromis sans pour autant laisser tout passer. C'est ce que l'Union européenne a fait, le 22 mars dernier, en décidant de sanctions contre la Chine sur le dossier ouïghour, alors même que nous discutons de l'accord d'investissement. Comme je l'ai dit, la diplomatie est l'art de l'équilibre ; c'est aussi celui de la désescalade. Dans ces conditions, il me semble- autant que faire se peut -que nous devrions trouver un juste milieu en activant les dispositions qui permettent d'associer Taïwan, en tant qu'entité, aux grandes organisations sans pour autant engendrer de provocations. à ce stade, le groupe du RDSE estime qu'il faut encore laisser du temps à la diplomatie et aux discussions. Un temps nécessairement plus long que celui du Parlement. C'est pourquoi nous ne prendrons pas part au vote.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de résolution nous invite à soutenir la décision du Gouvernement d'appuyer le retour de Taïwan au sein de l'Organisation mondiale de la santé, son entrée à l'Organisation de l'aviation civile internationale, ainsi que dans la Convention des Nations unies contre la corruption et Interpol, dans un contexte de pressions internationales importantes de quelques pays. L'île, qui, pour rappel, a joui du statut de membre observateur de l'OMS de 2009 à 2016, n'a plus été invitée par l'organisation onusienne depuis l'élection à sa tête de l'indépendantiste Tsai Ing-wen. Ing-wen. Le problème qui semblerait se poser aujourd'hui est de savoir sous quelle forme se ferait le retour de Taïwan ... En tant que région rattachée à la Chine ou en tant que pays souverain ? Sans même s'interroger sur les revendications territoriales de l'île ? En 1964, la France avait su se distinguer des autres pays occidentaux en reconnaissant diplomatiquement la République populaire de Chine et en entretenant des relations privilégiées avec Pékin. sept ans avant que l'Organisation des Nations unies ne reconnaisse la République populaire de Chine et lui réserve le siège au Conseil de sécurité occupé depuis 1950 par Taïwan. Des relations parfois difficiles, certes, mais tout de même suffisamment suivies pour que Paris fasse office d'interlocuteur exigeant et respecté. Il convient de rappeler la participation de Taïwan sous la dénomination « Taipei-Chine » à de grands événements internationaux comme les jeux Olympiques et Paralympiques ou à des instances multilatérales

Il est vrai que Taïwan, de fait, existe et dispose d'un organe législatif, exécutif et administratif. De plus, le renouvellement des générations renforce la distance prise avec Pékin. En effet, 85,6 % des Taïwanais sont nés après la séparation de l'île et du continent. Cependant, je me permets de rappeler que, sur cette île, la Constitution de la République de Chine est toujours applicable et intègre dans son territoire la Chine continentale et des territoires russes, indiens ou encore mongols. Le contexte de confrontation déclenchée par Donald Trump est stratégique, politique et commercial. Ce contexte n'est d'ailleurs pas étranger au regain des mobilisations sur Taïwan, à l'enjeu de la rivalité stratégique. Toutefois, nous ne pouvons pas omettre non plus que la situation actuelle laisse craindre une escalade pékinoise qui pourrait aboutir à un conflit. Que gagnera la France à s'impliquer dans cette stratégie de confrontation ? La réponse occidentale doit-elle être de mettre de l'huile sur le feu ou d'apaiser la situation ? Cette proposition de résolution, malheureusement, s'inscrit par ailleurs dans un alignement inquiétant de la France dans la roue des États-Unis. Son siège au Conseil de sécurité de l'ONU mais aussi son histoire avec Pékin lui donnent pourtant la responsabilité de se placer en conciliatrice. Les exemples du GATT ou du Comité international olympique montrent qu'un espace existe, d'autant plus que l'île et le continent sont particulièrement dépendants. L'adoption d'une telle proposition de résolution serait-elle de nature à aplanir les tensions ou, au contraire, à les exacerber jusqu'à un point de non-retour ? Au vu des réactions officielles de Pékin, on peut craindre une rupture franco-chinoise, qui à bien des égards Soutenir cette proposition de résolution serait s'inscrire dans l'agenda stratégique porté par les États-Unis et sortirait la France de sa position de neutralité dans le dossier. C'est pourquoi notre groupe s'abstiendra. La

Madame la présidente, mes chers collègues, le 1 janvier 2020, à Wuhan, en Chine, le docteur Li Wenliang de l'hôpital central était incarcéré avec sept de ses collègues. Deux jours plus tôt, il avait lancé l'alerte sur le fait que sept personnes travaillant sur le marché aux animaux de la ville avaient contracté un virus proche du SRAS. Le docteur Li Wenliang a été contraint de reconnaître qu'il perturbait l'ordre social. Le 7 février 2020, il comptera parmi les premiers Fort de son expérience du SRAS en 2003, Taïwan a su anticiper l'épidémie. Dès le 31 décembre 2019, elle alertait l'OMS sur la possibilité d'une transmission interhumaine du virus apparu à Wuhan. Elle n'a pas été entendue. Il faudra attendre le 20 janvier 2020 pour que Pékin se résigne à reconnaître que le virus était transmissible entre humains, date à laquelle l'OMS a qualifié la situation « d'urgence de santé publique de portée internationale Nous savons aujourd'hui que ces trois semaines perdues en janvier ont eu des conséquences tragiques pour la planète. La mise à l'écart de Taïwan des réflexions et actions conduites par l'OMS nuit aux intérêts de la communauté internationale. C'est précisément ce qui apparaît dans l'exposé des motifs de la proposition de résolution que nous présentent aujourd'hui nos collègues Alain Richard et Joël Guerriau, que je remercie chaleureusement. Le 20 février 2020, je déposais une question écrite interrogeant notre gouvernement sur les initiatives qu'il pourrait prendre afin d'intégrer Taïwan dans les discussions internationales sur le nouveau coronavirus. Des milliers de Français vivent à Taïwan ; je voulais éviter que ces compatriotes se retrouvent en dehors de la protection de l'OMS. Ce 20 février, le monde dénombrait alors 2 012 morts du covid, dont 2 008 en Chine, un à Hong Kong, un à Taïwan et un en France. Un mois plus tard, le 31 mars 2020, avec quatre-vingt-quatre parlementaires, nous cosignions une tribune appelant à l'intégration de Taïwan au sein de l'OMS, sur l'initiative de notre collègue André Gattolin. L'épidémie s'est répandue sur la planète, rebondit avec ses variants- britannique, brésilien, maintenant indien. Les ravages se poursuivent. Le 20 février 2020, Taïwan comptait vingt-trois cas de covid et, je vous l'ai dit, un seul décès. À ce jour, l'île totalise 1 121 cas confirmés et seulement douze décès, pour 23 millions d'habitants. Taïwan est le territoire qui compte le moins de cas et de décès recensés dans le monde. Dès l'origine de l'épidémie, l'industrie taïwanaise a produit 13 millions de masques par jour. Résultat : pas de confinement et une vie sociale, scolaire et économique qui se poursuit normalement, mais sous précautions. En juin 2020, en réponse à ma question écrite posée quatre mois plus tôt, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, m'indiquait qu'il souhaitait que Taïwan puisse être associée aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé afin d'éviter de créer un vide sanitaire. Force est de constater que, depuis, rien n'a changé. Taïwan ne sera même pas conviée en tant que membre observateur de la prochaine assemblée générale de l'OMS de nombreuses organisations internationales. Voilà pourquoi il nous est apparu, au sein du groupe d'échanges et d'études avec Taïwan, présidé par notre collègue Alain Richard, que l'heure était venue de déposer une proposition de résolution en faveur de l'association de Taïwan aux travaux de plusieurs organisations internationales. l'île est également exclue d'Interpol, ce qui crée des brèches considérables à l'heure où elle fait partie intégrante de la mondialisation et joue un rôle majeur dans la lutte contre les criminalités transnationales. Taïwan n'est également plus en mesure de participer à l'OACI, alors qu'elle en a été membre fondateur et qu'elle occupe une position clé pour le transport et le contrôle aériens en mer de Chine. En matière d'environnement, enfin, Taïwan ne peut pas participer aux réunions de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et ce bien que la société taïwanaise soit à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique. Tous ceux qui nous écoutent doivent s'interroger : pourquoi Taïwan ne fait naturellement pas partie de l'OMS, d'Interpol, de l'OACI et de tant d'autres instances de coopération internationale ? Comment en sommes-nous arrivés là ? La réponse se trouve de l'autre côté du détroit : la dictature du parti communiste chinois n'aime pas le régime démocratique en place à Taïwan. Malgré l'animosité entretenue par le régime communiste de Pékin, la société taïwanaise s'est émancipée dans le progrès, la liberté d'expression et les valeurs démocratiques occidentales. L'évolution de la société taïwanaise, affranchie et connectée, avec un pouvoir d'achat équivalent aux régions les plus développées du monde, ne peut être compatible avec les pratiques du régime totalitaire chinois, dont le « système de répression institutionnalisé » à l'encontre des musulmans ouïghours dans la région du Xinjiang révolte le monde. Comme nous, les Taïwanais observent avec effroi l'emprise du régime de Pékin sur tout le peuple chinois un contrôle de masse, un contrôle de chaque instant que les nouvelles technologies permettent de perfectionner à l'infini, au point de vous retirer toute intimité. Le pourcentage d'individus se définissant comme taïwanais est passé de 17,6 % en 1992 à 67 % en 2020, avec une progression de 10 % l'an passé. En octobre 1989, à l'occasion d'une visite en RDA, Mikhaïl Gorbatchev déclarait à son homologue est-allemand, ardent opposant aux réformes, « celui qui est en retard sur l'histoire est puni par la vie ». Quelques semaines plus tard, le mur de Berlin tombait. En clamant que Taïwan est une province intégrante de son pays, Xi Jinping est en retard sur l'histoire ! Taïwan, c'est un quart du PIB de la France. Avec 110 postes diplomatiques répartis dans 75 pays, c'est le trente et unième réseau diplomatique mondial, devançant des pays comme la Suède ou Israël. C'est la vingtième armée du monde, à niveau équivalent du Canada. L'île est souveraine. Taïwan est indépendante de fait. Certains diplomates soucieux de plaire à Pékin disent : « Moins on parlera de Taïwan, mieux cela vaudra. » Je pense tout le contraire.

puissance commerciale et onzième économie la plus libre du monde, Taïwan agit conformément aux conventions des Nations unies sur les droits de l'homme. En matière de démocratie, elle en a fait autant que n'importe quel autre pays pour faire avancer l'égalité. L'ONU a été créée pour les êtres humains. Je vous le demande, mes chers collègues, pourquoi l'universalité des droits de l'homme proclamée par les Nations unies ne s'appliquerait pas à Taïwan et à ses 23 millions d'habitants ? « Unissons-nous dans une pensée commune, et répétez avec moi ce cri : Vive la liberté universelle ! », lançait Victor Hugo. En débattant de cette proposition de résolution, au moment où, à Londres, le G7 déclare dans un communiqué son soutien affirmé à la participation de Taïwan aux organisations internationales comme l'OMS, nous envoyons un signal fort à nos alliés, à tous les peuples libres du monde.

le jour où la Chine s'éveillera à la démocratie, la Chine sera Taïwan ! Bravo ! Excellent

Je souhaite profiter de ce débat pour élargir mon propos à la problématique de Taïwan sur la scène internationale. Après de longues années de bienveillance au nom d'un prétendu « partenariat stratégique », la diplomatie européenne commence à à ouvrir les yeux sur la réalité chinoise. La crise du covid, bien sûr, mais aussi la répression de Hong Kong et des Ouïghours ont accéléré ce réveil de l'Europe. Alors qu'elle était restée jusqu'alors très mesurée dans ses réponses aux provocations chinoises, elle commence enfin à hausser le ton. Sa nouvelle stratégie sur la zone indopacifique et ses nouveaux projets de coopération avec l'Inde et l'Australie vont dans le bon sens, celui d'une lucidité sur la réalité chinoise. à mon tour la suspension par la Commission européenne, voilà deux jours, des négociations en cours sur l'accord d'investissement global entre l'Union européenne et la Chine. Alors que la Chine remet en cause les intérêts économiques européens et qu'elle n'hésite pas à poursuivre son travail de proximité avec certains pays certains pays d'Europe centrale et orientale pour essayer de les détacher de la solidarité européenne, la prudence concernant Taïwan n'est plus de mise. Aujourd'hui, Pékin s'éloigne manifestement d'une résolution pacifique, et le Président Xi se montre de plus en plus menaçant. À cet égard, l'omission des termes « réunification pacifique » dans le discours de mai 2020 du Premier ministre chinois à l'Assemblée nationale populaire ne fut pas accidentelle. Outre ses déclarations agressives, la Chine multiplie les manoeuvres militaires, maritimes notamment, et l'armée chinoise pratique l'escalade, aussi bien par l'ampleur manoeuvres qu'en termes d'incursion spatiale en mer de Chine méridionale. Cela ne signifie pas que la guerre sera déclenchée demain, mais une chose est sûre : la Chine se comporte comme si elle s'y préparait. La puissance navale chinoise augmente, celle des États-Unis diminue. C'est la première fois depuis la chute de l'Union soviétique qu'une grande puissance est en mesure de rivaliser avec l'US Navy. Certes, les États-Unis ont commencé à réagir avec un plan de réarmement naval massif, mais, dans les simulations opérationnelles, ils semblent avoir de plus en plus de mal à pouvoir s'opposer militairement à une opération chinoise contre Taïwan. De façon plus générale, et avec tous ses défauts, l'horrible Donald Trump a eu au moins un mérite : il a ouvert les yeux de l'Amérique, et les nôtres sur la réalité de la menace chinoise, menace économique et commerciale, bien sûr, mais aussi diplomatique et de plus en plus militaire. Je reprendrai le parallèle de notre collègue Cadic, en comparant Taïwan des années 2000 à Berlin des années 1950. Pendant la guerre froide, Berlin avait une signification symbolique forte, mais ce n'était qu'un symbole ; en plus de sa portée symbolique, Taïwan a une véritable valeur économique et stratégique.

Face à la Chine, mes chers collègues, la naïveté n'est donc plus permise, et, nous le savons tous, la pusillanimité ne mène à rien, sauf à l'impuissance. Soyons lucides : la Chine est un régime fort, qui ne respecte que la force et qui ne croit qu'aux rapports de force. Face à de tels régimes, on sait d'expérience, hélas, où conduit l'esprit munichois. Quand on croit éviter la guerre au prix du déshonneur, on finit toujours par avoir et la guerre et le déshonneur. Alors, certes, personne ne veut la guerre avec la Chine, mais, si nous voulons sauver l'honneur, il faut soutenir Taïwan. C'est pourquoi nous devons soutenir la participation de Taïwan- démocratie exemplaire -à toutes les organisations multilatérales et voter la proposition de résolution qui nous est soumise. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je me réjouis que cette proposition de résolution sur Taïwan ait été inscrite à l'ordre du jour de notre assemblée. Je m'en réjouis d'autant plus que j'avais déposé une question écrite sur cette thématique en janvier 2020. C'était, autant que je le sache, la toute première question sur le sujet, plusieurs autres ayant été déposées ensuite sur le même thème par mes collègues de l'Assemblée nationale et du Sénat, dont certains se sont exprimés précédemment. Outre une demande d'état des lieux sur les excellentes relations bilatérales entre nos deux pays, je m'interrogeais sur le bien-fondé de l'isolement imposé à Taïwan depuis la résolution 2758 de 1971, alors même que Taïwan, sous la direction de la Présidente Tsai Ing-wen, est un modèle de démocratie, applique à la lettre les recommandations de l'ONU, a un comportement et un bilan exemplaires- notamment en matière de protection de l'environnement, d'énergie verte, de soins médicaux, d'éducation, de lutte contre la pauvreté un PIB équivalent à celui de la France ou du Japon et un taux d'alphabétisation de 98,7 %. J'y indiquais également qu'à l'heure de l'apparition en Chine de virus rappelant le SRAS de 2003- ma question, j'y insiste, a été publiée en janvier 2020 -, une participation de Taïwan à l'OMS, ne serait-ce qu'avec un simple statut d'observateur, pouvait s'avérer très utile pour aider à juguler les risques d'épidémie. Le jour même où je déposais ma question au Sénat, ce 20 janvier 2020, l'OMS se décidait enfin à qualifier l'épidémie de covid d'« urgence de santé publique de portée internationale mois plus tard, au regard des douze décès dus au covid-19 à Taïwan depuis le début de la pandémie, sur une population de près de 24 millions d'habitants, on ne peut que déplorer que la voix de Taïwan, voix de l'expérience, de la science et de la sagesse n'ait pas été entendue.

Aujourd'hui même, un laboratoire taïwanais a annoncé avoir mis au point un vaccin contre l'entérovirus 71, efficace notamment chez les enfants de moins de six ans et qui pourrait être extrêmement utile à toute l'Asie.

Mais cette année encore, Taïwan ne sera pas représentée au sein de l'Assemblée mondiale de la santé qui se tiendra à la fin de ce mois à Genève. Ce n'est pas tolérable, d'autant d'autant moins que Taïwan avait été acceptée comme observateur à l'OMS de 2009 à 2016 et que refuser la participation de Taïwan à cette organisation, au regard des 150 millions de cas de covid aujourd'hui dans le monde et des 3,5 millions de morts, serait criminel. Si la France a toujours tenu une même position d'ouverture, le ministre Le Drian me répondant en 2020, ainsi qu'à tous ceux qui avaient posé les mêmes questions par la suite, que la France était favorable à la participation de Taïwan aux organisations internationales quand cette participation répondait aux intérêts de la communauté internationale- c'est le cas pour l'OMS -, la voix de la France est restée quelque peu isolée. Il est donc de notre devoir, bien sûr, d'appuyer cette démarche. Aujourd'hui, la situation commence à évoluer. Ainsi, le G7 réuni à Londres a annoncé, hier, dans sa déclaration des ministres des affaires étrangères et du développement, son souhait que Taïwan puisse participer de manière significative au Forum de l'OMS et de l'Assemblée mondiale de la santé, car «

contraindre Taïwan à un isolement diplomatique et multiplie les déclarations agressives, voire les menaces. Certains nous ont même conseillé d'être prudents pour éviter les foudres du pays et de son représentant à Paris, qui ne s'est pas privé, dans un passé récent, d'abreuver d'insultes les parlementaires français. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous laisser intimider.

comme l'est d'ailleurs Taïwan. La diplomatie est l'art de la prudence, du compromis et des tout petits pas. Nous ne saurions attendre de la France qu'elle avance seule contre ses propres intérêts économiques. Il serait trop facile d'agiter les bras pour faire des effets à cette tribune, et je m'en je pense vraiment que ce serait tout à l'honneur de ce grand pays qu'est la Chine et de ce grand peuple de 1,4 milliard d'habitants de faire preuve de magnanimité et de respecter les plus petits que

voisin. Les avancées et les richesses de Taïwan, avec un PIB en prévision de croissance de 4,6 % pour 2021- près de 8,2 % de plus au premier trimestre par rapport à l'année dernière -, ses innovations technologiques et sa politique industrielle dynamique peuvent susciter envies, appétits,

; oui, la Chine se réarme. Mais je crois profondément que l'honneur d'un parlementaire, c'est aussi de savoir faire preuve de courage et d'affirmer haut et fort ses convictions. Alors, oui, madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je veux le dire haut et fort : c'est notre devoir d'aider Taïwan à retrouver la place que ce pays mérite sur la scène internationale. L'équilibre géopolitique mondial implique que nous soutenions Taïwan, car, pour que nous puissions atteindre une paix, même relative, sur notre planète, pour que nous puissions travailler enfin à l'amélioration du climat, de la sécurité, des conditions de vie des citoyens du monde dans leur ensemble, nous devons développer notre coopération internationale et, surtout, nous devons inclure tous les acteurs dans les organisations internationales. Pour nous, parlementaires, c'est aussi une question de courage. Alors, oui, mes chers collègues, ayons le courage d'aller de l'avant, ayons le courage de ne pas nous laisser intimider par les gesticulations et les invectives, ayons le courage de dire ce que nous pensons être juste. Renforcer nos partenariats en matière sanitaire et médicale est indispensable, mais Taïwan doit aussi avoir le droit de participer à toutes les organisations internationales où son expertise pourrait être utile. Je pense notamment à Interpol, à l'Organisation internationale de l'aviation civile, au débat sur le climat. Je voudrais aussi dire à tous ceux qui, ici ou ailleurs, auraient la tentation de Munich qu'on ne respecte jamais un adversaire qui s'aplatit, mais que l'on craint et respecte celui qui, même s'il sait qu'il ne gagnera pas, a le courage de se battre pour ses convictions lorsqu'il les sait justes. Je souhaiterais aussi m'adresser à mes amis chinois, parce que, nous le savons, ils nous écoutent ou ils nous liront. Mais de quoi avez-vous peur ? Vous êtes un grand, vous êtes un magnifique pays, vous n'avez rien à craindre de Taïwan, qui ne veut que la paix Vous avez tout à gagner, au contraire, d'une coopération pacifique dans l'intérêt de vos peuples. Alors, s'il vous plaît, aidez Taïwan à vous aider, aidez-nous à vous aider, aidez-les à vous aider, ne serait-ce qu'en matière médicale Parlez-leur, écoutez-les, et le monde n'en sera que meilleur : il sera plus sûr, plus stable. Et c'est aussi votre intérêt, c'est l'intérêt de la Chine dans son ensemble.

La démocratie taïwanaise se construit à l'ombre de la Chine. Situé à moins de 200 kilomètres des côtes chinoises, ce territoire de près de 24 millions d'habitants dispose de son propre drapeau, de son hymne, de sa langue, de ses institutions judiciaires et de son Parlement, mais n'est reconnu que par seize pays et connaît un isolement diplomatique croissant.

d'autant que Taïwan représente un modèle d'acteur responsable dans de nombreux domaines, par exemple la lutte contre le changement climatique, comme le montre son adhésion aux principes fixés par la COP21. Les progrès scientifiques de Taïwan en matière de technologies vertes sont remarquables et méritent d'être reconnus, tout comme son centre national des technologies et des sciences pour la prévention des sinistres, que nous avons visité. partenaire solide dans les domaines économique et de sécurité, et les plus de 2 300 Français qui y vivent dynamisent nos relations commerciales et nos actions de coopération. Enfin, la loi sur le mariage pour tous, votée en mai 2019, ou la « révolution des tournesols », menée en 2014 par les jeunes étudiants du numérique contre l'ingérence chinoise, sont des marqueurs d'une démocratie bien vivante. Son succès réside également dans sa gestion de l'épidémie de la covid-19. Taïwan, cela a été rappelé, a été le premier pays à prévenir l'Organisation mondiale de la santé des dangers d'une contamination humaine, alors même que ce pays reste exclu de cette organisation. Dans sa réponse à mon courrier du 18 mars 2020, le ministre Le Drian précisait que la France soutenait la participation de Taïwan aux travaux de l'OMS et de l'Assemblée mondiale de la santé, une reconnaissance de fait de sa maîtrise exceptionnelle de la crise sanitaire. En effet, sa gestion épidémique est un modèle pour le monde entier. Le système de traçage a été consenti par la population sans obligation étatique. Cette responsabilisation collective alliée à la présence de masques chirurgicaux, à des quatorzaines ciblées et à un système de santé performant a permis de maîtriser très vite la diffusion du virus. Le pays n'a pas eu recours à un seul confinement ni couvre-feu et n'a pas mis son économie à l'arrêt. Cette efficacité a aussi été rendue possible grâce à la transparence et à la confiante participation de la population dans sa gestion de la crise. Un exemple dont nous pourrions d'ailleurs utilement nous inspirer chers collègues, vous l'aurez compris, le partage de son expérience et sa contribution ne peuvent qu'être bénéfiques à la communauté internationale dans tous les domaines cités par les auteurs de cette proposition de résolution, Alain Richard et Joël Guerriau. Comme l'a annoncé mon collègue André Vallini, tous les membres de notre groupe voteront cette proposition de résolution, pour que la France apporte un soutien clair à l'intégration de Taïwan au sein des instances internationales. La parole

cette proposition de résolution en faveur de l'association de Taïwan aux travaux de plusieurs organisations internationales, présentée par Alain Richard, Joël Guerriau et nombre d'entre vous ici présents, que je ne saurais tous citer. C'est un moment effectivement utile utile et important. Vous connaissez la politique constante de la France sur la question de Taïwan : elle reconnaît le gouvernement de la République populaire de Chine comme seul représentant de la Chine depuis 1964 et n'entretient pas de relations diplomatiques avec Taïwan. Cependant, la France développe des coopérations avec ce pays dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler « la politique d'une seule Chine ». Elle considère en outre que les relations entre les deux rives doivent reposer sur un dialogue constructif, dans la mesure où il est dans l'intérêt de tous que la voie du dialogue soit privilégiée, afin que la paix et la stabilité puissent être préservées dans le détroit de Taïwan. Des échanges dynamiques, des coopérations riches se développent entre nos deux territoires, qui font de Taïwan un partenaire important de la France en Asie. Vous avez été nombreux à signaler la place dans l'économie mondiale de l'île- vingt et unième économie mondiale -, sa place dans les chaînes de valeur mondiales, en particulier dans l'industrie

Cette coopération tient compte aussi de la vitalité de la société civile taïwanaise, vous l'avez relevé les uns et les autres, de la remarquable réussite de la transition démocratique de l'île initiée dans les années 1980. Taïwan accueille de surcroît une importante communauté française, évaluée à 4 000 personnes, qui font l'objet d'une attention de tous les instants de notre part. À travers en particulier le bureau français de Taipei et le bureau de représentation de Taipei en France, la France et Taïwan entretiennent et développent des échanges soutenus dans les domaines économique, industriel, scientifique, de l'innovation et de la technologie, mais également en matière culturelle culturelle et éducative. Nous partageons avec l'île des valeurs démocratiques, une ambition commune pour la promotion des droits de l'homme. D'ailleurs, notre ambassadeur pour les droits de l'homme s'y est rendu en janvier 2020. En matière culturelle, la France et Taïwan entendent poursuivre et approfondir leurs coopérations déjà très denses. Taïwan fait partie des trente-sept territoires identifiés en 2019 par le ministère comme prioritaires pour l'export des industries culturelles et créatives françaises. J'ajoute que la coopération éducative et universitaire a pris une tournure significative : le nombre d'étudiants français à Taïwan a tout simplement

Taïwan. Bien que n'étant aujourd'hui reconnue sur le plan diplomatique que par quinze États, l'île développe une politique active sur la scène internationale, y compris auprès des pays avec lesquels elle n'entretient pas de relations diplomatiques. Parallèlement, Taïwan est membre d'une trentaine d'organisations intergouvernementales ; j'évoquais l'OMC, mais on pourrait citer l'APEC, la Banque asiatique de développement et tant d'autres. Elle participe, en tant qu'observateur ou membre associé, aux travaux d'une vingtaine d'organisations intergouvernementales ou d'organes subsidiaires ; je pense à l'OCDE, à la BERD ou à la Banque interaméricaine de développement.

favorables lorsque le statut des organisations le permet et que cette participation répond aux intérêts objectifs de la communauté internationale. Il y a donc là une convergence très claire. C'est manifestement le cas pour les organisations internationales que vous avez citées dans la proposition de résolution : l'OMS, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, mais également l'OACI, Interpol. Je crois que la pandémie de covid rappelle chaque jour, cruellement, depuis plus d'un an, que la santé des femmes et des hommes du monde entier requiert l'engagement et la coopération. Sans la coopération, nous ne vaincrons pas cette épidémie. Il en est de même pour les questions climatiques, pour les transports, pour la sécurité soit nous réussissons ensemble, soit nous échouons ensemble. Cela appelle donc une réponse collective. S'agissant plus spécifiquement de la santé mondiale, puisque nous sommes à quelques jours de cette réunion importante à l'OMS, les chiffres parlent d'eux-mêmes Taïwan a remarquablement contenu l'épidémie. C'est pourquoi sa contribution et le partage de son expérience sont essentiels à l'ensemble de la communauté internationale, à l'heure où il faut oeuvrer collectivement. Vous avez rappelé les uns et les autres les chiffres : douze morts seulement sur une population de plus de 23 millions d'habitants. Indéniablement, Taïwan a su tirer tous les enseignements de l'épidémie de SRAS en 2003 pour réagir rapidement et efficacement dès les premiers signes d'apparition de la maladie. Nous n'oublions pas qu'au printemps 2020 Taïwan a fait don d'équipements médicaux- masques, appareils respiratoires -à plusieurs de ses partenaires dans le monde, dont l'Union européenne et la France. Jean-Yves Le Drian, qui, hélas ! ne pouvait être présent aujourd'hui dans l'hémicycle- il est au Liban -, a eu l'occasion de dire lui-même, en novembre dernier, que nous étions favorables à ce que Taïwan participe aux réunions de plusieurs organismes internationaux, dont l'OMS, car il est essentiel que tous les acteurs qui

pour que Taïwan soit associée aux travaux de l'OMS. Nous le ferons à titre national, nous l'encourageons au niveau européen, nous l'avons fait encore il y a quelques jours avec nos partenaires du G7. Compte tenu de ces différents éléments, permettez-moi de souligner que la proposition de résolution portée par les membres du groupe d'échanges et d'études Sénat-Taïwan, sous votre conduite, monsieur le président Richard, présente de réelles convergences avec la position du Gouvernement que je viens d'exprimer. Je salue ici l'esprit constructif de votre initiative. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, la France ne veut pas que la question de la participation de Taïwan aux organisations internationales devienne un enjeu politique. L'enjeu est tout autre : répondre aux intérêts objectifs de la communauté internationale. C'est dans cet esprit que la France soutient cette participation de Taïwan aux organisations internationales lorsque leurs statuts le permettent. le souligne à nouveau : le fonctionnement optimal de ces organisations appelle une approche inclusive, condition d'un multilatéralisme efficace pour apporter des solutions aux grands défis de notre monde. Au-delà de l'examen de cette proposition de résolution, vous me permettrez, puisque le sujet est au coeur des travaux de votre groupe d'études, monsieur le président Richard, de souligner que nous suivons de façon extrêmement précise l'évolution de la situation dans le détroit de Taïwan. Nous avons noté à cet égard que les incursions militaires dans la zone d'identification et de défense aérienne de Taïwan se sont multipliées depuis l'an dernier, jusqu'à devenir presque quotidiennes. Je le redis : la stabilité dans le détroit est essentielle pour la sécurité de la région ; c'est la raison pour laquelle nous réprouvons toute tentative de remise en cause du de même de même que toute action susceptible de provoquer un incident et de conduire à une escalade dans le détroit. Je crois pouvoir vous dire que nous partageons cette préoccupation avec l'ensemble de nos partenaires de l'Union européenne.